la parole est à Madame Laure Darcos ce, pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, merci Monsieur le Président, je souhaitais faire la mise au point suivante sur les scrutins publics numéro 38 et 41 ma collègue Christina plus j'souhaité voter pour. Merci, cher collègue, acte est donné de cette mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyste politique des scrutins. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour 2023. Dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'article 32 quater avec un amendement 82, monsieur le rapporteur, un amendement de la commission. Oui, bon, merci monsieur le Président, bonjour à tous, oui, donc l'amendement propose la suppression d'une demande de rapport. C'est un rapport qui étaient sollicités pour encadrer les activités financières, immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits elle pèse épargnants à cet article alors déjà, faisons en sorte que l'article puisse s'appliquer et donc qu'on fera un moment à la doctrine du Sénat, c'est une demande de de donc, c'est une demande Merci monsieur le Président, bonjour à tous, mesdames et messieurs les les sénateurs donc cette. Rapport effectivement qui a été introduit dans la loi, par un amendement à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'en remet donc à la sagesse de votre assemblée. Merci donc je mais aux voix l'amendement de la commission de suppression avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté, et donc l'article est supprimé le 32 qu'inquiet, amendement 83 83 ce rapporteur. Oui, de nouveau, une demande de rapport donc un amendement de suppression, là c'est un rapport concernant la compensation des révélations salariale dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, c'est un vrai sujet intéressant mais ça fait partie également des missions de la CNSA, donc c'est une demande de suppression.

Il était adopté l'article 32 sexy est que l'amendement 84. Une demande de suppression d'un rapport sur les aides à l'investissement, voilà donc voilà conformément.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, donc l'article L 313 Tiret 12 Tiret de, dans sa rédaction actuelle laisse trop de place à interprétation et plusieurs autorités s'en saisisse pour refuser de conclure des contrats de compétence conjointe, les établissements particulièrement visé par ce type de pratiques étant les femmes et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés aussi cet amendement propose qu'en cas de compétence conjointe, il ne puisse être conclu qu'un seul contrat pour les établissements et services concernés. Merci, monsieur le rapporteur. C'est le président, alors certains établissements sont placés sous l'autorité d'un plusieurs tutelles et c'est le cas notamment des femmes, c'est le cas des sommes par exemple, la législation actuelle donc autorisé la pluralité de contrats cet amendement propose un seul contrat en cas de compétence conjointe d'ailleurs, c'est ce qui se pratique dans certains départements, sans support juridique clair en accord entre la RS et et les conseils départementaux et je vous rappelle, c'est une préconisation du rapport réalisé par mes soins, au nom de la casse sur la simplification des politiques publiques dans le du handicap sera un avis favorable. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs je vous confirme effectivement que cette possibilité est déjà ouverte dans les départements, mais que cette obligation risquerait néanmoins de bloquer la signature de certains contrats Henri édifiant trop le le processus cette disposition par ailleurs constituerait en outre un cavalier social donc, le gouvernement est défavorable à cet amendement. Merci donc je le mets aux voix avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté, nous passons l'article 33, une prise de parole de Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le le président je profite ici de cet article 33, la réforme du financement des services de soins à domicile pour dire quelques mots sur une disposition adoptée lors de la LF SS 2020 et qui pour nous est emblématique des maux de notre système actuel, en effet, l'article 34 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2020 a entièrement transformé le système de financement actuel des établissements assurer une activité de psychiatrie en introduisant une dose de T2A 2 Abssi est appelé tarification de compartiments et de c'est pour les intimes, on ne connaît que trop les effets pervers et destructeur de la T2A dans les hôpitaux publics pour ne pas s'inquiéter de ses effets sur la psychiatrie ce genre de financement favorise la recherche d'actes rentables et les indicateurs retenus nous inquiète, le nombre d'actes de journée de demi-journées, la durée du séjour, la file active la qualité de codage, l'âge des patients, et de nombreux professionnels en pédopsychiatrie et psychiatrie ne cesse de nous alerter ces indicateurs vont orienter automatiquement les pratiques vers des actes qui permettent de recevoir, de très nombreux patients au détriment du temps nécessaire à leur à leur consacrer consultation ponctuelles, programme de courte durée, bilan divers prescription de médicaments, toutes et tous s'inquiètent du devenir des personnes qui ont besoin de soins attentifs relationnel pluridisciplinaire au long cours ajusté au plus près de leurs besoins, toutes ces procédures, à l'inverse de ce qu'il faut faire, sont l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, les soignants craque et dénonce un système qui les empêchent de la Coupe d'accomplir leur mission, parlant de perte de sens de leur métier, nous avions déposé un amendement déclarée recevable, c'est très regrettable, car pour nous, il est urgent de revenir sur cette réforme de financement qui est inadapté à la conception du soin psychique, Merci, cher collègue, je mais au voilà l'article 33 qui est pour. Qui est pour l'article 33 qui est contre. Qui s'abstient, il était adopté l'article 33 bis 2 amendements identiques, le 539 Monsieur Savary. merci Monsieur le Président, les dispositions votées à l'Assemblée nationale, vise la forfaitisation de la pas et si les départements partagent l'objectif de proposer un accompagnement aussi approprié que possible aux besoins des personnes âgées, il convient aussi de prendre en considération les incidents sur les Budgets départementaux et la nécessité de ne pas que l'on complexifier la gestion administrative des dossiers, c'est d'ailleurs pour cette raison que la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit la possibilité de forfaitisée là, pas à condition qu'un contrat pluri-et objectifs des moyens souhaite élaboré par ailleurs départements de France, rappelle que les départements n'ont pas été consultés sur cette modification majeure, semble-t-il, en conséquence, il demande que ces dispositions ne soit pas votée dans l'immédiat, afin d'engager les réflexions nécessaires ou, à défaut de les proposer au département qui le souhaiteraient, sans que cela soit une obligation. la forfaitisation va dans le sens d'un accompagnement aussi approprié que possible des personnes âgées en permettant de moduler cette prise en fonction des besoins, le temps de la concertation souhaitée par notre collègue nous est donné par le renvoi des conditions des aides forfaitisation à un décret,

qui oblige quelque part une concertation avec les départements qui n'a pas eu lieu pour l'instant, et donc à ce titre-je vais demander : demande de retrait pour ces 2 amendements au bénéfice des amendements 1000 100 42 1000 100 43 qui auront sécurisé les relations entre l'État, les départements, pardon, mais avant d'autres transporteurs. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs, je me permets une prise de parole développé pour à la fois vous présenter l'article et l'amendement du gouvernement. Qui propose de le reformuler, vous le savez, les plans d'aide humaine à la à l'allocation personnalisée d'autonomie ou plan d'aide à pas sont aujourd'hui fixés sur une base mensuelle actuellement les heures non utilisés sur un mois, sont perdus pour le bénéficiaire, on sait pourtant que des événements ponctuels tels qu'une hospitalisation, une absence de solution alternative conduit souvent à ce que ces heures ne soit pas utilisé et qu'en même temps les situations comme le retour d'hospitalisation peuvent-elles au contraire créer un besoin plus important, la question de l'assouplissement de la règle en vigueur se poser donc et vos homologues de l'Assemblée nationale ont souhaité avancer dans ce sens, je partage cette préoccupation qui renvoie à la question du libre choix par les bénéficiaires à l'accueil, à laquelle je suis très attaché, la mesure retenue par l'Assemblée nationale prévoyait une forfaitisation de la Pac, il n'allait pas sans poser de difficultés pratiques concrètes tant pour les gestionnaires que pour les départements et même pour les bénéficiaires, c'est pourquoi l'alternative qui vous est proposé vise à s'affranchir du cadre autant pour elle mensuel en ouvrant la possibilité de reporter les heures non consommés sur six mois pour mieux tenir compte des besoins des personnes sans remettre en cause la personne de l'évaluation mensuelle des besoins ni les modalités de calcul de la participation des personnes, c'est le moyen qui est déjà utilisée actuellement pour la PCH depuis la loi de 2020, visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap que le rapporteur mouillé connaît évidemment bien la disposition permis ainsi une convergence entre les 2 prestation dans un domaine où elle est pertinente : un décret précisera en préciserait les modalités et un temps de concertation avec les départements que nous avons également consulter et le représentant des services d'aide à domicile doit être ménagé, c'est pourquoi il vous est proposé une entrée en vigueur en 2024 pour qu'on puisse avoir le temps de de cette concertation, et j'insiste sur ce point qui répond, des jeux d'ores et déjà à la préoccupation de certains d'entre vous, que vous venez d'émettre et qui sera évidemment central dans les travaux à engager. Donc c'est un avis défavorable pour les amendements de suppression donc je, je l'ai mais aux voix ces deux amendements de suppression de 500 pardon Monsieur Savary. Non, je crois que le rapporteur a demandé de retirer les amendements si mes collègues sont d'accord, donc je pense qu'il est plus judicieux de les retirer et surtout après les explications et je ferai des commentaires dans les amendements sur. 539 et retiré, donc le 591 retiré aussi donc les deux amendements sont retirés l'amendement du gouvernement été présenté et donc on a des sous-amendements, le 842 monsieur Leno. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur a été clair dans son explication : monsieur le Ministre, vient de s'exprimer aussi, il s'agit dans cet amendement, d'imposer la vie des des départements, je vous remercie. Merci, mais 143 c'est identique, il est défendu monsieur rapporteur donc. Oui, monsieur, j'ai déjà donné des explications donc favorable sur l'amendement 1122 sous-amendé par le 1142 ou 1143 donc, elle avait favorable pour les trois.

Simplement, Monsieur le Ministre, bon c'est un amendement qui est si j'ai bien compris comme ça un article bis qui a été rajoutée à l'Assemblée nationale.

parce que c'est au détriment des personnes suivies et des personnes âgées, parce qu'on voyait, hein, comme les finances ne sont pas extensibles que peuvent faire les départements, je ne dis pas qu'ils le font, c'est compte tenu d'un coup plus cher, on fait moins d'heures l'hôtel il y a moins de service de rendu à la population, et puis la modifier complètement le calcul, ça m'arrange différents critères, alors ça peut être tout à fait intéressant puisque la personne est avait effectivement une autonomie qui qui évolue, il n'empêche que ce type d'approche différente mérite une concertation large et c'est ensemble, à ce moment-là que les choses peuvent bouger éventuellement au département de de faire des propositions, suivi par le ministère derrière quand elles sont tout à fait acceptable, ce que je dis pas de façon à ce qu'elle soit bien comprise par toutes et tous. Oui merci monsieur le président, il me semble que des départements peuvent très bien faire remporter les heures, moi il me semble que le enfin il ne sont pas je suis sûr que le Rhône, la fait la métropole de de Lyon la garder, c'est-à-dire que les effectivement ce que vous proposez n'importe quel département peu de façon autonome, le faire déjà voté voter un article, là, dans le cadre du conseil départemental pour le faire, donc voilà, c'était juste pour dire à leurs soit on on le rend obligatoire, ça peut être un objet d'amendements, mais en tout état de cause, aucun département n'est privé de de pouvoir établir ce report possible sur six mois voire sur l'année civile. Chers collègues, donc je mets aux voix les deux sous-amendements identiques 1142143 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés et je mais aux voix l'amendement 1122 du gouvernement ainsi sous- amendé avec un avis favorable de la commission. Qui est pour, Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je mais on voir l'article 34. Qui est pour, Qui est compte qui s'abstient-il être adopté même vote pour le 33 quater même vote il est adopté au 33 qu'Quiès on vote aussi même bottes adopté 33 sexy une prise de parole de Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le le président le 14 mars 2018 les députés. Monique Iborra et Caroline Fiat remettaient leur rapport sur la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Epad depuis les constats sont toujours les mêmes, toujours aussi accablant et, bien sûr, nous avons tous en tête le scandale Orpea mais je dirai de manière un petit peu familière, c'est l'arbre qui cache la forêt, qu'il s'agisse d'une volonté de profit de la part des actionnaires ou d'une insuffisance des dotations dans les EPHAD public le manque de personnel est criant et il génère de la maltraitance institutionnelle, la souffrance des résidentes et des résidents, mais également des soignants est aujourd'hui en quelque sorte la norme résidents qui reste des heures dans leurs excréments par faute de temps ou de moyens toilettes en moins de 6 minutes sur des corps qui sont souvent fatigués et meurtris, malnutrition, soins dentaires quasi inexistant personnes alitées 24 heures sur vingt-quatre sans même changer de position, ce qui entraîne des escarres qui ne sont pas toujours soigné en fait, c'est une situation qui est très alarmante qui n'est pas bien, bien sûr, mais quand même qui est très normatives en quelque sorte et les familles oscillent entre angoisse et culpabilité et on voit là des raisons pour lesquelles beaucoup de soignante change de profession, elles ont des troubles musculo-squelettiques des il y a beaucoup d'accidents de travail à répétition, hein, c'est supérieur au aux travaux aux aux accidents qu'il y a dans le bâtiment et des épuisement professionnel, or cette situation dramatique est aggravé par le développement des Epad privées à but lucratif, comme l'a montré, donc le scandale Orpea et on voit bien que dans les EPHAD public il y a aussi des situations qui sont très lourdes, d'où l'importance d'encadrer absolument les choses et surtout d'embaucher du personnel, il faut que la norme s'assoit un personnel pour un résident et on en ligne, on est loin de ce compte-là, je vous remercie. Alors, de nouveau, nous sommes dans une demande de rapport concernant notamment l'instauration d'un ratio minimal d'accord autrement. Des résidents par du personnel soignant, alors c'est un sujet extrêmement important, on a vu que c'est une référence dans tous nos débats, quoi qu'il arrive, je ne suis pas certain que le rapport soit nécessaire puisque, il suffit de reprendre déjà les rapports existant, je pense notamment à celui de la Cour des comptes qui fixe clairement des seuils, donc, de nouveau, c'était l'avis défavorable. Sachez, non c'est pas un avis défavorable, c'est une demande de suppression monsieur mais sagesse du Gouvernement sagesse donc je, je, mais oh vous pardon madame Cohen. je comprends hein le l'intervention de de notre collègue Philippe mouiller, c'est sûr que je crois que on on est toutes et tous, bien au fait de la situation donc faire un énième rapport n'apporterait pas grand chose je partage, mais Monsieur le le ministre, j'aimerais quand même que vous puissiez même si vous avez émis un avis de sagesse, vous puissiez devant devant nous ce matin, vous vous engagez à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnel dans les les en vous ayez l'engagement d'avoir entendu finalement ben là, les plaintes, les plaintes à la fois des soignants, des résidentes et des résidents mais également également des familles, alors j'ai cru comprendre que vous étiez attentif à cette situation et que vous alliez suivre ça de manière très précise, mais plus que des intentions, peut être que ce matin, c'est l'occasion pour nous d'entendre les engagements concrets parce que le personnel s'en allant, hé bien il y a besoin d'embauche et donc il a besoin d'améliorer leurs conditions de travail, quel est votre plan à ce sujet, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Savary. Oui, juste pour rappeler qu'effectivement il y a des difficultés dans les EPHAD mais aussi des pas dans lequel ça se passe bien quoi, il faut quand même pas jeter complètement, le ratio par personnel c'est effectivement insuffisant mais il y a aussi cette motivation du personnel qui est déterminante, on sait que le personnel est motivé et que les personnes âgées ne sont pas toutes maltraité parce qu'on a quand même encore besoin d'une structure correspondant à des Epad soyons attentifs à cela, je ne me permettait de le rappeler. enfin comme comme René-Paul Savary je pense qu'il faut qu'on fasse attention de pas jeter l'opprobre sur l'ensemble d'un secteur vous avez précisé que ça ne se passait pas comme ça dans tous les Ehpad mais c'est quand même important aussi de souligner que la grande majorité des Epad fonctionne de façon plutôt satisfaisante, avec des personnels qui sont extrêmement engagés et dont, je, je tiens à souligner l'engagement dans ce PLFSS on prend les choses en main, on s'engage sur la trajectoire de recrutement de 50000 professionnels soignants dans les 5 prochaines années on langage avec les trois mille et vous savez que alors je sais que plusieurs de de vos collègues qu'on aille plus vite, néanmoins, vous savez que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir recruter des personnels qui soient formés, il faut les attirer, il faut les former, il faut les fidéliser et donc c'est pour ça que le CNR bien vieillir comporte un axe complet qui est portée par Myriam El Khomri, qui a déjà beaucoup travaillé sur ces sujets-là, sur la question des métiers et on importera d'ailleurs un focus, pas seulement sur les Epad mais aussi sur le travail à domicile parce qu'on connaît aujourd'hui les difficultés de nos intervenantes à domicile et donc c'est bien l'ensemble de ces mesures qui vont permet de renforcer l'attractivité des métiers, je me suis engagé également et je le précise, à renouveler la stratégie sur de lutte contre la maltraitance d'ici à la fin de l'année, j'ai saisi également 3 corps d'inspection pour pouvoir pour pouvoir alimenter cette cette stratégie et ça fera partie des éléments qui, j'en suis persuadé rendront plus attractifs, nous Epad et rendront la qualité et la sécurité dans ses épate beaucoup plus fort. monsieur le président, oui, je voulais rebondir sur les propos de mon collègue René-Paul Savary, on a parlé Madame Cohen, les troubles musculo-squelettiques, il y a aussi beaucoup de l'établissement qui investissent dans des rails au plafond pour aider à porter les malades qui font des des formations justement pour arriver à porter, donc moi aussi je voudrais pas qu'on mette tous les ait pas dans le même dans le même panier, il y en a où ça se passe mal, mais il y en a aussi beaucoup, ça se passe bien, et je vous tenez aussi à le souligner, merci. 91 la Commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, donc, l'article est supprimé, article 35 inquiète le 92, monsieur le rapporteur. on continue dans les demandes de rapport, donc là, de nouveau, c'est un amendement de suppression d'un rapport qui pour évaluer le coût sur les comptes publics et sociaux de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée en établissements pour personnes âgées, voilà, donc bon, très bien, c'est, c'est un sujet intéressant mais de nouveau, je ne suis pas certain que ça suscite un rapport. Sagesse ça du gouvernement Madame Cohen. Je veux remercier Monsieur le Ministre, pour sa réponse parce qu'il a été très attentif à mes propos, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas dit que tous les Epad entraînait une maltraitance institutionnelle, loin s'en faut, et heureusement, donc c'est clair, en tout cas, il y a au moins un, une personne présente, qui l'a entendu la la la question effectivement de l'embauche, c'est un tout petit pas, Monsieur le Ministre, parce que vous savez que toutes les organisations syndicales demandent et les personnels et collectifs 100000 embauches par an sur 3 ans, c'est-à-dire 300000 et nous avons fait le calcul : 170 millions d'euros pour recruter dans les EPHAD ça représente un demi-poste de un demi-poste de plus dans chacun des 7000 Epad donc voilà, c'est un tout petit pas, c'est mieux que rien, mais il est, il faudrait en faire un plus grand voilà je vous remercie. Merci je mais aux voix l'amendement 87 de la commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'article est supprimé l'amendement adopté et après c'est à cet article le deux amendements le 372 Monsieur Madame Procaccia ou Monsieur Beulin. Monsieur Balland, allez-y. Merci Monsieur le Président, cet amendement vise à demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi, évaluant le coût de l'instauration d'un forfait prévention santé visuelle ce forfait permettrait au préventeur de santé visuelle de se rendre au domicile des patients sans reste à charge pour ces dossiers vous avez évidemment un certain nombre d'arguments qui vous sont présentés à la suite de cet amendement, les chutes sont responsables chaque année d'au moins 130000 hospitalisations la vision et donc l'un des cinq risque ayant à Shutter identifié voilà pourquoi cet amendement a été

co-signataire pour ce sujet important dans la prévention santé visuelle alors juste avant, on vient de supprimer un rapport qui demandait la même chose l'propose de réintroduire, donc je vous propose un avis défavorable sur cet amendement. Merci, monsieur le Ministre.

au même titre que les troupes de l'audition et de la nutrition, ainsi que la peur de la chute que la que l'inactivité et l'inadaptation logement tout d'abord le gouvernement partage comme vous l'importance de la santé visuelle, notamment chez les personnes âgées pour qui la baisse d'acuité visuelle peut entraîner des chutes et favoriser la perte d'autonomie, c'est pourquoi, dans le cadre du plan anti-chute des personnes âgées 2022 2024, le gouvernement prévoit de renforcer les actions portées sur l'ensemble des facteurs de chutes, dont les troupes de la vision, le présent Plfss prévoit la mise en place de rendez vous de prévention à différents âges clés de la vie, dont 65 65 ans, et 70 ans, les troupes de la vision pourront donc y trouver une place de choix, enfin nous engageons également les travaux de définition de repères spécifique pour le dépistage des troubles de la vision associées au vieillissement presbytie glaucome, cataracte en effectuant une nouvelle saisine de la Haute autorité de santé pour l'inscrire au sein de son programme de travail pour toutes ces raisons je suis défavorable à votre amendement. Il retiré merci le 608 monsieur Fiole R. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, la 5ème, branche pour être pleinement effective doit s'accompagner d'une véritable politique de soutien à l'autonomie et permettent une réelle amélioration des droits des personnes en situation de handicap ou âgées, quelle que soit leur âge et leur projet de vie, pour cela, elle doit impérativement répondre aux besoins croissants de financement, or, si le rapport Libault à dresser un constat précis des besoins de financement pour prévenir et soutenir la perte d'autonomie des personnes âgées, il existe peu de données sur le financement public nécessaire pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes en situation de handicap pour garantir une politique de soutien à l'autonomie à la hauteur, il est urgent de mieux évaluer les besoins de financement supplémentaires pour assurer l'autonomie de ces personnes, mais aussi de leurs familles et proches ses dents aussi cet amendement de notre collègue Artano demande au gouvernement un rapport estimant les besoins des adultes et enfants en situation de handicap ainsi que les moyens financiers supplémentaires à dégager. Et monsieur le rapporteur. Monsieur le président, alors je vous qu'en première lecture, lorsque j'ai vu l'amendement j'ai longuement hésité avant d'appliquer la doctrine sénatoriales et donc ce serait une demande de retraite, pourquoi, parce que c'est vrai que le point que vous évoquez est essentiel puisque ça fait des mois, des années que nous sollicitons une véritable évaluation des besoins dans le domaine du handicap aujourd'hui, qu'est ce que l'on voit, on a des briques, on a des bouts d'information, on a des départs devront par département, mais aujourd'hui on est, on est capable de dresser, je dirai, la liste des possibilités de l'offre, mais en matière de besoins, on a aucune évaluation c'est vrai dans le médico-social, c'est vrai en matière d'emploi c'est même vrai en matière d'éducation ayant en tête que, même pour la rentrée scolaire, on est incapable d'évaluer les besoins d'accompagnement des enfants en situation d'handicap pour les différents, je dirais, types de handicap concernés, donc on voit bien qu'il y a un vrai problème d'observatoire du des besoins, j'avais d'ailleurs moi-même proposé en tant que rapporteur, un amendement pour la mise en place d'un observatoire qui a été donc rejeté, auteur de l'article 40 et donc ce point essentiel alors si moi ça me semble court, parce que quand je vois où actuellement les les travaux qui sont enclenchées, vous avez tout à l'heure, nous aurons un amendement du gouvernement qui propose justement de je dirais de, de, de doter la CNSA d'outils complémentaire en matière d'informatique voilà donc moi ce que je vous propose, c'est de retirer cet amendement mais je me tourne vers la porte de la la commission affaires sociales du Sénat parce que je pense, c'est une vraie mission que nous pourrions porter toujours l'évaluation des besoins ont conjointement avec la CNSA et les départements qui ont une vision assez précise également la situation voilà donc demande de retrait, mais le sujet est tellement, tellement important et tellement nécessaire dans ce dans ce où on fait finalement une politique publique sans outil de pilotage, donc c'est un peu compliqué et donc je me tourne vers la prendre la commission sociales pour solliciter une mission. Sur ce sujet, donc nous avons de retraits Alors Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre : avis défavorable du gouvernement pour des raisons similaires merci madame Nadar. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, juste une précision pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur le rapporteur, dans chaque département, avant chaque rentrée scolaire, on pourrait quand même commencer à faire des réunions communes entre les MDPH et l'éducation nationale, ce qui ne se fait pas de manière naturelle et c'est pour ça qu'on manque, aider à ESH et que les les enfants se retrouvent sans suivi dans les écoles. Merci Monsieur Savary. Oui, moi je partageais propos du rapporteur et si Madame la présidente de la commission, on était d'accord, ça peut être un travail d'évaluation déjà des financements par l'Amex il y avait besoin, hein, moi je suis prêt à ce qu'on lance là de façon à ce qu'on fasse un état des lieux, ce qui aidera quand même par rapport à cette 5ème, branche à éclaircir un un petit peu les tuyauteries budgétaire notamment, ce qui est important quand même. Merci madame Meunier. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, moi je souris un peu intérieurement aux propos de notre rapporteur Philippe mouiller parce que il reconnaît la l'impératif de d'un un d'un vrai travail sur ce sujet dont on parle depuis des années ici, et en même temps ils refusent le travail par le l'amendement de notre collègue filières qui exactement dans le même sens, donc je ne vois pas pourquoi on refuserait un travail parlementaire et nous on on serait prêt à y travailler au sein de la commission des affaires sociales, donc si notre collègue ne retire pas groupe socialiste votera l'amendement présenté par Monsieur. Madame la présidente de gauche. Oui merci monsieur le président, nous on refuse pas un travail parlementaire on refuse un rapport que le gouvernement de remettre dans six mois dans les 6 mois qui suivent la loi c'est pas tout à fait pareil quand on voit le succès des rapports ou l'an dernier, concernant notre commission sur 22 rapport demandé et encore on avait tout supprimé tous ceux du Sénat pratiquement, donc je dis : on a eu un qui a été remis, donc quand même, mais en même temps, faut pas rêver, en demandant des rapports qui n'arrive jamais, en revanche, je suis tout à fait favorable, on en avait déjà parlé il y a quelque temps avec Philippe mouiller et on verra comment on s'organise entre La Mecque, c'est la commission pour faire ce travail. Merci monsieur Fiole écoutez, monsieur le président, si j'ai bien entendu l'engagement de la présidente de la commission a mené cette mission je retire le le dossier. Merci donc il le 608 et nous passons à l'article 34 Monsieur. merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est au nom de de Valérie Létard que j'interviens sur cet article, bien évidemment, il s'agit pas de remettre en cause les deux heures par semaine de soutien nécessaire pour les bénéficiaires et les personnels des Saad, que ce soit pour les objectifs ou pour les questions plutôt de perte d'autonomie ou de repérage des fragilités, nous partageons cet objectif d'autant plus, il y a un véritable enjeu qui consiste à empêcher la baisse de la qualité des stades, mais évidemment, la question est celle du du financement

c'est un débat essentiel puisque, aujourd'hui, dans le nord 80 pour 100 du financement de la pas et portée par le département, c'était 50 % à à la création et donc pour toutes ces raisons, nous posons la question Monsieur le Ministre, de financement de de ces deux heures sans remettre bien et on vous dit évidemment en cause, le sens de cette mesure et et son utilité, je vous remercie. Merci, chers collègues, l'amendement 540 Monsieur Savary.

cependant tous les n'est officiel de la pas ont pas forcément besoin de ces 2 heures de vie sociale par semaine, dans la mesure où elles bénéficient ces personnes d'un soutien familial sans faille ou profite encore d'une vie sociale active. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de préciser qu'il s'agit d'une possibilité, autrement dit qu'il revient à l'équipe médico-social de proposer ce temps dédié selon les besoins de la personne et avec l'avis de la personne, et ce pour 2 raisons : la première, et que l'équipe sur le thé, les équipes sur le terrain sont les mieux à même de cibler les personnes qui en auront le plus besoin, sans qu'il s'agisse forcément de tous les bénéficiaires de la la seconde est d'une question de moyens humains et financiers, un compte rapide pour un département de près de 300000 habitants cela nécessiterait 446 ETP en plus dans les alors que, actuellement, il y a déjà des difficultés énormes de recrutement, c'est la raison pour laquelle il semble raisonnable que la possibilité soit introduite à travers cette mesure. Si Monsieur rapporteur. Alors sur cet amendement dont j'entends l'argumentaire porté par Monsieur Savary, mais ce serait une demande de retrait parce qu'aura la rédaction de l'article est déjà clair et donc votre demande est satisfaite puisqu'on dit l'équipe propose donc ça veut dire que de leur qu'on propose, ce n'est pas une obligation, et c'est bien l'équipe pluridisciplinaire qui fera des propositions autour de tout cela mais je profite de ces prises de parole en complément de de la vie pour rebondir sur l'intervention de Monsieur Annaud et la question du financement parce que même si je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours entre le l'État et les départements, donc ça peut être l'occasion au cours de votre avis, Monsieur le Ministre, de nous de répondre à la question posée par Monsieur Leno donc un avis demande de retrait. Merci, monsieur le Ministre, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs. J'ai effectivement répondre à et nous, que je remercie d'ailleurs d'avoir salué la l'intérêt de cette mesure, qui je vous le rappelle, est une pro, une promesse du président de la République d'augmenter les. Les plans d'aide ah pas de deux heures une, une mesure qui va à la fois. Améliorer les plans d'accompagnement des des personnes pour permettre de renforcer du lien social réhumaniser aussi les interventions des des aides à domicile et, ce faisant, permettre aussi, hé bien d'améliorer l'organisation des du travail des intervenantes à domicile donc répondant en partie à votre préoccupation monsieur le le sénateur Savary vous dire qu'effectivement concernant les départements, j'ai mis en place depuis un mois environ, un comité des financeurs qui s'est déjà réuni plusieurs fois, qui a permis d'aboutir d'ailleurs vous verrez tout à l'heure je vous présenterai un amendement du gouvernement pour pouvoir concrétiser les accords que nous avons pu obtenir à l'occasion de ces 2 dernières réunions avec les départements, l'idée étant de mettre en place une méthode de travail qui permettent à la fois d'assurer d'assurer un dialogue et une concertation des départements avant que nous puissions prendre des décisions et à inscrire dans la loi un certain nombre de de mesures comme celle-ci, on a prévu cette cette concertation précisément pour ces 2 heures en repoussant à 2024 la mise en oeuvre de de de ces deux heures et donc on parlera pratique comment les mettre en oeuvre et s'assurer effectivement que ça permettra d'augmenter les plans d'aide, mais surtout de ne pas mettre en difficulté des départements pour revenir sur la situation particulière du Nord, j'en ai déjà discuté effectivement avec la sénatrice Valérie Létard et avec le président Poiret, on sera extrêmement attentif avec la CNSA évidemment à s'assurer de la qualité de ce dialogue et de ne pas mettre les départs. Moment en difficulté quant à l'amendement avis défavorable également du du du gouvernement pour les mêmes raisons que que le rapporteur. Puisque ces heures ne sont pas obligatoires que elles feront l'objet d'une évaluation des besoins, avant d'être attribués, le cas échéant, et que par ailleurs je vous l'ai dit concernant l'attractivité des métiers, les difficultés de de recrutement, elle vise précisément à renforcer et améliorer l'organisation du travail des intervenantes à domicile. Merci, monsieur le Ministre, Madame Jouanno. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, moi je salue cette nouvelle disposition, cependant je pense qu'il faut être très très vigilant sur le financement pour les départements parce qu'il y a effectivement des territoires où il y a beaucoup de personnes qu'il faut soutenir et puis je voudrais dire que c'est une question importante pour les aides à domicile, pourquoi, parce que justement les aides à domicile, se plaignait très souvent d'exécuter un certain nombre de tâches très rapidement, il n'avait pas à ce moment de de lien social avec les personnes, donc ça c'est une très belle avancée, je voudrais dire aussi que c'est une belle avancée pour les personnes âgées, cependant il faut regarder pour chacune d'entre elles, où en est le plan d'aide parce que quand on est au plafond, justement, hé bien on ne peut pas profiter de deux, heures supplémentaires, ou alors c'est au détriment des heures qui sont déjà effectués, donc, sur ce point là, il faut être très attentif, d'autant plus que l'année dernière avec l'augmentation hou la la la, revalorisation des salaires dans ce domaine, on est arrivé à moins d'heures pour certaines personnes âgées donc vigilance, c'est un petit pas pour plus d'humanité, mais il faut être vigilant mais. c'est une mesure tout à fait certes intéressante parce que la convivialité, pour moi, c'est une mesure de prévention ah Inde notamment de troubles cognitifs derrière, donc ça veut dire que c'est valable, bien entendu, pour les personnes à domicile. Parce qu'elles sont particulièrement isolées, notamment en milieu rural, et quand la famille est éloignée, donc c'est intéressant mais quand ces personnes vont dans une autre structure un établissement d'autonomie intermédiaire ou un habitat inclusif ou bien Nepad, il ne faut pas que cette mesure soit supprimé, ça veut dire que, elle continuera, elle devra porter aussi bien sur la pas à domicile que là-bas, on n'est pas largement qui fait que on doit recalculer l'ensemble derrière, surtout si on veut forfaitisée derrière la pas ça refait un calcul, donc soyons attentifs à cela, c'est un élément nouveau et c'est surtout qu'il faudra mettre en face de ça, des moyens importants, très importants, hein, c'est la raison pour laquelle il faut véritablement compte tenu que c'est cette mesure est sur le compte des départements, faire en sorte qu'il soit particulièrement associé à l'évolution des choses me semble-t-il, donc, Monsieur le Président. Oui, je voudrais dire, voilà le 540 et retirer nous passons 2 amendements identiques, le 512 madame Meunier. Merci monsieur le président, j'ai écouté attentivement les propos du ministre et c'est vrai qu'ils vont dans le bon sens, mais cet amendement précise encore en tout cas, souhaite préciser encore ce qu'on entend par lien social et l'amendement propose de remplacer cette notion par participation à la vie sociale, ce qui ferait que vous savez que dans le domaine du handicap, cela déclenche cette notion de participation à la vie sociale, un besoin d'aide humaine et en la matière, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous déplacer pour aller au cinéma, faire ses courses ou toute autre activité à l'extérieur quand on est en en en dépendance, donc, cet amendement vise aussi à connaître, Monsieur le Ministre, vos intentions concernant, hé bien cette fameuse barrière d'âge hein, les bénéficiaires de la PCH aide humaine et les bénéficiaires de la pas en ce qui concerne les personnes âgées donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur vos intentions merci. Et ici 120 identique Madame Lottin il est défendu il il est défendu, je voudrais juste m'a apporté une toute petite enfin pas une précision mais vraiment insister sur le fait que ces 2 heures de de lien social, enfin peu importe la manière dont on les appelle va permettre aussi de faire sortir un petit peu les, les contingents d'heures qui sont très souvent beaucoup trop limité pour une aide à la toilette avec des des personnels qui sont hyper pressés dont le travail et le maintien à domicile est rendu difficile, donc moi je salue la mesure et puis effectivement la. Merci, monsieur le rapporteur. rapporteur. Le président, alors c'est une évolution rédactionnelle qui est proposé, mais au-delà de l'évolution rédactionnelle, c'est un vrai débat vrai sujet qui le débat de la période âge et quelque part le rapprochement a pas PCH, c'était un sujet que que nous y portons depuis déjà qu'avait plusieurs mois et donc qui renvoie aussi à la problématique de tout à l'heure des besoins, analyse des besoins des évolutions, le reste à charge, la prise en charge, voilà, donc ça c'est un point important, mais on ne peut pas enlever cette thématique là de du débat de la relation entre l'État, les départements parce que de nouveau la question derrière c'est : qui finance quoi et quelle prix charge raisonnable peut être porté alors de cette rédaction différente, quelque part, c'est un signe, c'est un qui est donné et les associations du monde handicap ont réagi suite au dépôt de cet amendement plutôt négativement parce que modifié quelque part est enclenché ce cette cette évolution

qui doit être mis sur la table qui dans tous les cas, doit être traité en corollaire des sujets que nous avons évoqués d'une vision globale, finalement de l'évolution des politiques publiques en matière de handicap, donc une demande de retrait pour ces 2 amendements, monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Meunier je confirme effectivement que c'est un sujet qu'on a sur la table aujourd'hui de discussions notamment avec les départements pour pouvoir traiter de cette approche globale de l'autonomie et ça fait longtemps que vous discutez, je le sais, du rapprochement entre la paille la PCH, ça me semble un peu prématuré aujourd'hui de, de, de vous apporter une réponse parce que ça nécessite des discussions importantes tant d'ailleurs d'un point de vue philosophique du point de vue du du coup aussi de ces mesures et de la répartition des, des, des charges et donc ça fait partie des sujets qu'on qu'on discutera dans le temps. Avec les départements et la CNSA pour revenir à vous amendement et le rapprochement entre l'appellation de ces 2 heures de. Convivialité et celles existant dans le cas de la PCH de participation à la vie sociale, ces 2 dispositifs si elle vise à favoriser le maintien du lien social ne s'exerce pas tout à fait de la même façon, selon les mêmes modalités le dispositif de la PCH vise à permettre aux personnes de sortir de chez elle pour participer à des activités extérieures et donc ainsi s'inclure dans la société, la spécificité du temps de du temps dédié au lien social prévu dans l'appart et que cette au domicile de la personne qu'il intervient et non dans un lieu extérieur 16 heures serviront à repérer aussi les fragilités et à prévenir l'isolement social comme on l'a dit leur instauration vise aussi à améliorer les conditions de travail des auxiliaires de vie, je le redis, en limitant le fractionnement de leurs interventions, il en augmentant leur temps de travail, donc les objectifs des 2 dispositifs sont clairement distincts, je suis donc défavorable à votre amendement qui rapprocherait les de dénomination. Revient pas sur l'argumentation de l'objet de cet amendement, puisque je l'ai fait dans la prise de parole, je voulais juste définir l'objet, il s'agit de relever la part du financement de la CNSA ah la, pas de 7 70 % à à puisque ce déploiement efficient immédiat de la mesure notamment permettrait de dépasser de 0,4 % la cible visée par le gouvernement dans le projet de loi et il permettrait un soutien renforcé de la CNSA au département en matière d'appât, je vous remercie, merci monsieur le rapporteur. donc, donc, cet amendement propose quelque part un meilleur financement pour les départements, donc ça c'est une musique qu'on aime bien entendre ici dans cet hémicycle, voilà donc je vais mettre un avis favorable mais je voudrais surtout entendre Monsieur le Ministre, regarde de cette proposition parce que, de nouveau, on est dans les des débats, des négociations entre l'État, les départements essentiel voilà et donc pour une fois, on vous propose de modifier la participation avant même que vous augmentiez les charges ou en complément et donc je souhaite une belle initiative, donc celui année l'avis favorable sur cet amendement. Merci, monsieur le Ministre. C'est le président, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur. Sénateurs et nous. Comme vous le relevez l'article 34 prévoit bien d'augmenter la part des recettes de la CNSA dédié au concours à pas afin de financer la dépense supplémentaire induite par le nouveau dispositif d'accompagnement et de lien social, cette hausse des recettes de permettent de maintenir constante la part des dépenses couvertes par les recettes propres des départements puisqu'il s'agit de l'augmentation d'une charge relevant de la compétence des départements, par ailleurs, la dotation complémentaire visant à améliorer le service assuré par les services d'aide et d'accompagnement à domicile ou la dotation permettant au département de converger vers le tarif plancher sont pleinement des soutiens au département dans leur mission d'accompagnement des personnes âgées, plus largement, on pourrait évoquer une réflexion à mener sur sur les concours j'ai plaisir de vous dire que le gouvernement évidemment partage cette analyse, que nous avons commencé ce travail avec la CNSA sur une réforme des concours de la CNSA qui vise à compenser toutes ces mesures qu'on a inscrite au fil du temps dans les projets de loi de de financement de la Sécurité sociale notamment, et que ça fait partie du travail pour 2023 du comité des financeurs auquel je faisais référence tout à la tout à l'heure, donc de l'instance de dialogue entre l'État et les départements, et donc nous travaillerons dès le début d'année prochaine, c'est inscrit dans notre programme de travail sur cette réforme des concours des concours de la de la CNSA, qui est d'ailleurs inscrite, hein, je vous le rappelle dans la dans la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNSA, donc je suis défavorable à votre amendement. Merci Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Ministre, il y a les fonds puis la répartition des fonds : derrière hein alors moi je veux bien qu'on change un petit peu les différentes tuyauteries, mais moi je voulais attirer votre attention parce que quand on on on délègue des fonds à la CNSA qu'répartis après par contingentement on garde à chaque fois des fonds prudentielles on répartit pas tous les fronts, voilà donc on fait illusion des fonds condamne et puis comme les fonds prudentielles, on les a pas affecté, ben on prend une nouvelle mesure, et puis on dit bah, il reste un peu le fond prudentielles, donc on va la financer comme ça, c'est valable la première année, pas la deuxième, c'est de la cavalerie, ça veut dire qu'aussi, avec une recette, là aussi, on fait de dépenses.

on arrive à faire en sorte que l'argent n'est pas réparti, hein, et donc c'est là aussi au détriment de celui qui reçoit l'argent, à savoir le département pour en revenir à une et un rapprochement a pas PCH soyons attentifs, parce qu'on sait que cette PCH correspond derrière à des prestations fort différente selon le tien de handicap, hein, qui soient psychique ou notamment sensorielle avec les forfaits etc c'est pas forcément qu'le câble et ça générera automatiquement 2 des dépenses supplémentaires si ça répond bien aux préoccupations des personnes, pourquoi pas, mais si c'est par des rapprochements administratif et que ça ne correspond pas forcément à leurs préoccupations, je reste pour l'instant en observation par rapport à cette évolution. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, la difficulté pour l'ensemble des départements, c'est que nous avons des plans d'aide totalement différenciées d'un département à l'autre et que la part contributive de la CNSA n'est pas connu d'un département à l'autre l'autre et donc c'est vrai que, il y a tout ce qui est prudentiel et des discussions qui se font tout au long de l'année si le comité des financeurs que vous préconisez, je trouve que c'est une très bonne chose dès l'année prochaine, pouvait donner une lecture de l'ensemble des 101 départements sur la part contributive et versée pour des APA en fonction des territoires et en fonction du nombre de personnes âgées qui bénéficient de ces prestations d'APA, ça serait très bien, parce que sinon, chaque président discute après de manière l'uninominal avec son ministre de tutelle, par exemple, c'est le cas pour le département de la réunion qui demande à rencontrer le ministre de l'Outre-mer pour pouvoir discuter de l'augmentation éventuelle de sa part APA. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur.

qui est la complexité du système des tuyaux, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 13 tuyaux différents et si on voit l'évolution peut être passer à 16 tuyau différents dans la relation entre la CNSA les départements en matière de lisibilité, je pense qu'on peut mieux faire et même, même en matière de cohérence politique parce que des des politiques publiques, parce que c'est pas qu'à ce problème de versement, c'est un problème de vision globale et de et de cohérence voilà donc c'est aussi un message que l'on peut porter. Merci, monsieur le rapporteur je mais aux voix l'amendement 340 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je mais on voir l'article 34. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient il être adopté après cet article, 2 amendements identiques, le 137 Madame Miller. Oui, merci Monsieur le Président, 30000 établissements et services médico-sociaux existent aujourd'hui en France, autant de possibilités de soutenir les proches, les aidants de personnes accompagnées ou soigner au sein de ces établissements et services dans sa recommandation de bonnes pratiques professionnelles de 2015 le soutien des aidants non professionnels, la HAS proposé que les professionnels de ce secteur social et médico-social puisse soutenir les aidants de personnes âgées adultes handicapés ou souffrant de maladies chroniques, néanmoins, on constate l'impossibilité de la mettre en oeuvre, faute d'une clarification de ce public dans l'émission, des oeufs, SMS et de moyens alloués conseiller évaluer, orienter un projet aidant prend du temps et nécessite des compétences spécifiques, il est pourtant nécessaire de reconnaître le rôle et la plus value des SMS dans l'arsenal des solutions pour soutenir les aidants, en plus des dispositifs dédiés aux aidants, s'appuyant sur l'expertise d'une équipe pluridisciplinaire, ils peuvent faire l'interface entre les besoins du proche aidant et ceux de la personne aidée cette émission supplémentaire devant se traduire d'une part par l'ajout d'un Aléna cette à l'article L. 311 tirer un du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part par une dotation globale dont une partie sera forfaitaire pour pérenniser les actions dans le temps et une autre partie variable cette part vers variable sera déterminée en fonction de l'offre proposée l'ensemble des critères relatifs à la partie variable seront précisées par décret, je vous remercie. Oui, et donc je vais juste compléter je reprends beaucoup de de ce qui vient d'être dit cela quand même nécessite également des moyens supplémentaires qu'ils ne pourront ainsi être débloqués que si et seulement si, les missions des établissements sociaux et médico-sociaux vis-à-vis des proches aidants sont clairement établies dans le droit cet amendement se propose de mettre enfin en oeuvre les préconisations de la Haute autorité de santé et de permettre aux quelque 8 virgule 3 millions de proche aidant selon l'adresse de trouver un soutien auprès des 30000 établissements et services médico-sociaux avec lesquels la collaboration est essentielle : je vous remercie. C'est le président donc j'entends aujourd'hui les demandes situation de nos. Sénateurs à travers cet amendement est donc on ne peut qu'être favorable au fait de reconnaître le travail des aidants et de les accompagner, de les aider dans la révolution par contre votre amendement concerne l'intention donne quelques pas d'active aux établissements recommandations des des connaît son HS mais sans parler de financement puisque sinon ça article 40 et la difficulté, c'est qu'on demande un travail supplémentaire à des établissements et pourrait être bien souvent sur le terrain, certains petits établissements publics auront des difficultés sans dotation supplémentaire à assurer cette mission, donc le maître dans la loi sur les moyens, c'est un peu compliqué, on peut pas rester sur les intentions, donc ce sera une demande de retrait un argument supplémentaire, c'est que dans la logique de ce que nous avions évoqué l'année dernière au PLFSS nous avions mis en place, les centres de ressources et je pense que les centres de ressources dont le le experte dans des déploiements peuvent certainement intello si le débat de l'ensemble du territoire et donc des aidants, et donc pour l'instant les de ressources commence juste à se mettre en place, je pense que c'est un peu prématuré, je crois qu'il faut entendre le message, mais avant tout cas je serai défavorable à vos amendements pour les raisons évoquées. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices. Je vais essayer de vous montrer que votre amendement en réalité déjà satisfait puisque de nombreuses de SMS Conseil soutiennent oriente déjà les les aidants familiaux et les proches aidants cette mission peut être formalisée dans leur projet d'établissement et des moyens dédiés à ces actions peuvent être contractualisé dans le cadre des ses pommes signé avec les ARS ou les conseils départementaux le renouvellement de la stratégie en faveur des aidants, que j'ai annoncé lors de la journée nationale des aidants, le 6 octobre dernier intégrera les actions que peuvent conduire les oeufs SMS en soutien aux aidants, l'article que vous souhaitez modifier énonce les actions pouvant être mises en oeuvre par les établissements sociaux et médico-sociaux. La première mission énoncé à cet article recouvre déjà des noms des notions que vous souhaitez introduire dans votre amendement, votre amendement, me semble-t-il, n'est donc pas nécessaire et c'est pour cela que j'y suis défavorable.

Oui, monsieur le Président, en prolongement des engagements qui ont été pris par la la commission des affaires sociales, cet amendement donc rare que les dispositifs actuels de soutien de l'autonomie a pas et PCH sont insuffisants et trop parcellaires, et qui instaure par ailleurs des barrières dans l'accès aux droits, notamment en fonction de l'âge aussi, cet amendement propose de réfléchir à la crise à la création d'une prestation universelle d'autonomie, quelle que soit l'âge, l'état de santé ou le handicap qui permettent de garantir les moyens financiers d'une compensation intégrale effective et personnalisé sans exclusion d'aucune situation de de handicap, ce serait d'ailleurs en cohérence avec le caractère universel de la prise en charge et du soutien l'autonomie et avec la loi du 11 février 2005 qui prévoit la suppression des barrières d'âge en matière de compensation du handicap afin d'éviter toute rupture de droits. Merci, cher collègue de 934 Me Poncet Monge. Oui, merci Monsieur le Président, alors c'est une demande de rapport, mais j'aimerais quand même qu'on soit un peu attentif et que quelques fois on l'applique pas de façon aveugle, le refus du Sénat d'un d'un rapport car suite à la proposition de Michel Meunier suite au fait qu'on dit à moi suis débutatifs et caetera, il faut qu'on avance, j'entends ça, moi depuis 2 ans sur le la mise en oeuvre d'une prestation unique de compensation de l'autonomie. Parce que l'enjeu de l'égalité de traitement face au besoin d'aide et d'accompagnement à l'autonomie implique entre autres, entre autres mesures, la suppression de toute barrière d'âge, il s'agit, concrètement, de supprimer toutes les dispositions qui peuvent conduire à des ruptures ou à des différences d'accompagnement entre les personnes, comme l'avait mis en perspective le législateur à travers l'article 13 de la loi du 11 février 2005, quand même, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, or actuellement et en fonction de l'âge de survenue

l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire du secteur plaide de longue date pour l'abrogation des paris hier des barrières d'âge source d'inacceptables inégalités l'enjeu fondamental est celui de l'égalité de traitement de toute personne en risque de perte d'autonomie, quel que soit son âge, son projet de vie et se indépendant indépendamment indépendamment de son lieu de vie, supprimer la barrière d'âge permettra enfin de réduire le morcellement des dispositifs en sortant de la logique de catégorisation des publics et participera au changement de regard sur le vieillissement, notamment l'objet de cet amendement et de mesurer par une étude d'impact, enfin des hypothèses concrètes de la mise en oeuvre d'une prestation unique de compensation de la perte d'autonomie. Alors sur ces deux amendements, ça sera un avis défavorable puisque de nouveaux sur demande de rapport, simplement une précision pour l'amendement de Monsieur ah. éthanol 603 puisque là on parle de prestation universelle de tsunami, donc là on va au-delà du débat de la âge puisque le principe, là on est sur une compensation intégrale de l'ensemble des des besoins, donc on est déjà un degré supplémentaire, donc je vous pose déjà qu'on a elle fléchisse au débat des bavardages avant d'aller aussi loin, même si c'est un sujet qui est sur la table donc on est plus sur un rapport sur l'étude d'impact ou joue sur les mots, mais vous avez vu que la mission proposée par notamment notre commission devra réfléchir à tous ces éléments-là donc une demande de retraite. Monsieur le Ministre Mesdames, ma vie, mais ma vie Oui. C'est ce matin, je ai mais aux voix tout d'abord le 603 avec 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour 934 même vote il n'est pas adopté, nous passons 428 madame Jasmin. Merci monsieur le président, c'est un c'est un amendement de notre collègue plat qui concerne le non-recours à ASPA chez les personnes âgées de 65 ans, ce taux de ce taux de non-recours concerne la récupération sur la succession est très importante et dissuasive, démontre dénombrait en 2014 817000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, ce non recours sur succession concerne les familles très modestes des personnes retraitées, qui vivent dans des, dans des difficultés il y a une nécessaire de prendre en compte cette situation particulièrement pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, donc nous devons collectivement nous en parler de cette problématique pour améliorer les conditions de vie de ces personnes et tenter de trouver les meilleures solutions possibles merci. Si monsieur le rapporteur. Alors toujours une demande de rapport, mais cet amendement prévoit la donc la remise au Parlement d'un rapport. Sur les conséquences de mécanisme de récupération sur succession sur les taux de recours à la en outre-mer, notre collègue Cathy la potion a récemment rappelé dans ce rapport sur la proposition de loi tendant à assurer la revalorisation des pensions de retraite les plus faibles que le non-recours à l'espace semblé au principe même de récupération sur succession, source de défiance et au refus de certains bénéficiaires de faire appel à la solidarité nationale, qu'ils assimilent à l'aumône, c'est la question du niveau du seuil de récupération sur succession peut et doit être posée, son principe ne me paraît pas devoir être remis en cause, dans la mesure où certains bénéficiaires de l'ASPA justifie de faibles revenus, certes, mais dispose d'un Patrimoine important, il est logique que les montants versés de la solidarité nationale soit récupérer sur ce Patrimoine au décès de l'allocataire quoiqu'il en soit, au-delà de cet avis, ou en tout cas de ce contexte que je vous donne, c'est un avis défavorable.

vingt-quatre nous passons, article 34 bis Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, alors que la question de l'autonomie toute notre société, je crois que la question de la prise en charge et de là. L'accompagnement des personnes malades en situation de handicap ou de perte d'autonomie pose celle des conditions des aides qui sont mises en place et y compris celles des proches, mais au-delà, cette évolution, ainsi que le vieillissement de la population augmente la probabilité qu'un aidant familial accompagne plus d'une personne au cours de sa vie, chaque Français et Françaises et c'est souvent sur les femmes, qu'un que repose cette tâche aura l'occasion de devenir et aidant pour l'un de ses proches et se plusieurs fois au cours de sa vie, le congé de proche aidant existe mais il est imparfait dans sa durée dans son indemnisation, suscitant soit un un accompagnement soit, y compris des ruptures d'emploi, je crois qu'il est temps de réévaluer sa durée et son indemnisation pour qu'il soit réellement un droit opposable par les salariés, l'objet de cet article et d'évaluer l'application de l'article 54 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2 1000 22 et la subséquente opportunité d'élargir la durée, l'indemnisation du congé proche aidant, avant l'examen du projet Plfss si j'ai bien compris donc nous ne pouvons que qu'y souscrire je vous remercie. de nouveau demande de rapport donc un avis, donc là c'est une demande de suppression donc les concerne sur l'opportunité, Hergé la durée, l'indemnisation du congé de proche aidant qui est prévue cet article donc on demande une rapport alors que pour l'instant, on n'a pas encore voté l'Arctique, donc voilà demande de suppression de ce rapport. Sagesse. De la part du gouvernement donc je mais aux voix l'amendement 88 de suppression de la commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, et l'article supprimer l'article 34 terre un moment 89. De nouveaux demande de rapport donc donc on vous demande de supprimer ce rapport. Même avis, Monsieur le Ministre, même avis même vote. Le. Pardon madame Guy

depuis 2 ans, moi je me bats pour que l'extension de la JPA aux aidants de personnes atteintes d'un cancer puissent se faire trop de jeunes aidant, malheureusement aident un parent atteint d'un d'un d'un cancer, je pense que si le conjoint et dans pouvait obtenir le serait une belle avancée et ça permettrait surtout de soulager les familles et je trouve que, aujourd'hui, la JPA n'est pas adapté, c'est bien pour cela qu'il est si peut demander, je vous remercie. Qui est contre Qui s'abstient-il être adopté et donc l'article est supprimé, nous passons à l'article 35 amendement 731 Monsieur Iacovelli. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le passage du forfait habitat inclusif géré par l'ARS à l'aide à la vie partagée VP par les départements d'ici à 2025 est prévu depuis la loi de financement de la Sécurité sociale 2021, le passage à la VP permet un char, un changement, pardon de paradigme, car ce sont les personnes qui finance le projet de vie sociale et partager néanmoins la disparition progressive du forfait habitat inclusif n'est pas sans conséquences pour les porteurs de projets, le forfait étant sous forme de développement global versé au projet permettait une aide au démarrage les projets n'ayant pas de trésorerie font face à de nombreuses difficultés pour le démarrage du projet dans l'attente de connaître le montant du bénéfice de la VP si les habitants ne sont pas encore identifié et dans les discussions avec les financeurs qui demande une assurance de l'inscription du projet dans le dispositif de l'habitat inclusif et donc de la VP un maintien du forfait est à systématiser dans cette période de latence pour ne pas provoquer de fermeture de ses sites, compte tenu du fait que la CNSA massivement compenser le financement depuis 2021 de la VP, il apparaît nécessaire de maintenir le suivi du dispositif par la CNSA lorsque cette aide sera complètement décentralisée, merci l'objet de cet amendement, donc elle le maintien d'un forfait dans la période d'élaboration de démarrage des projets d'habitat inclusif, la mise en place d'ailleurs d'un bilan annuel réalisé par les départements, c'est un amendement essentiel car il corrige les difficultés engendrées par la création de la de la vie partagée notamment dans cette période particulière de transition, donc ça n'a eu favorable. Merci, monsieur le Ministre, dans les habitants inclusif, le concours a pour objet de financer une partie des dépenses des départements relatives à l'aide à la vue partagé, mais les coûts de démarrage des projets ne relève pas de la même de la aussi c'est la conférence des financeurs de l'habitat inclusif qui est l'instance au sein de laquelle les besoins d'aide au démarrage peuvent être discutées par ailleurs, un rapport d'évaluation de l'habitat inclusif et déjà élaboré chaque année au mois de juin par la conférence des financeurs de chaque département il est transmis chaque année à la CNSA et comprend des données relatives à la vie partagée au nombre et au profil des bénéficiaires, ainsi qu'à l'accès aux équipements chaque année un rapport synthétique et analytique et rédigé par la CNSA, sur la base de ces rapports afin de favoriser le développement de l'habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap pour ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement, il y a des fois, j'y serai défavorable. Merci, il est maintenu et est maintenu Monsieur Oui, merci, c'est un amendement fort pertinent cher collègue parce que on peut pas dire d'un côté, Monsieur le Ministre on est favorable à l'habitat inclusif et d'un autre côté, modifier une aide essentielle pour la transmettre derrière au département, hein. Parce que ce principe de l'État qui dit pour inciter une politique allait je finance à 100 % hou là à 80 % pendant un an, 2 ans, 3 ans et puis après, démerdez-vous, excusez-moi le terme, débrouillez-vous, je je retire, débrouillez-vous, il n'empêche que derrière, si les départements dans les, pas les moyens de suivre ça peut pas marcher, vous avez un objectif de 150000. Logement inclusif d'ici 2030, ça va pas tenir ce n'est pas possible : l'avantage de maintenir l'aide à l'investissement, c'est que vous pouvez lancer des projets sans avoir officiellement la liste des personnes qui vont rentrer dans ce type d'habitat, et c'est logique, on ne peut pas les connaître à l'avance et ses côtes la structure là qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont réservé le le logement que on peut ensuite montré le modèle et que les personnes du milieu environnant viennent dans la structure en conséquence faut impérativement trouver un système pour maintenir ça parce que je pense que l'habitat inclusif et vraiment l'intermédiaire entre le maintien à domicile à tout prix et, parfois, on laisse les personnes dans une situation d'isolement déplorable, hein, dans des fermes isolées, et cetera, loin de leur famille et les Ephad qui, derrière, sont d'une structure de plus en plus médicalisées qui sont en fait des, des, des, des hôpitaux pour personnes âgées, plus que des structures d'hébergement, compte tenu de l'évolution de l'âge et du vieillissement de la population, donc je pense, c'est tout à fait important de soutenir cet amendement.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs. Le système d'information harmoniser des MDPH repose actuellement sur la labellisation des systèmes d'information conforme à des exigences fonctionnelles attendu par la CNSA dans le contexte de la création de la 5ème, branche et du renforcement des attentes relatives à l'équité de traitement et à l'universalité des droits, ce modèle harmoniser atteint désormais ses limites et il est désormais proposé de basculer vers un système d'information unique pour Les MDPH la création de ce système d'information unique dont la maîtrise d'ouvrage est confié à la CNSA permettra d'offrir une plus grande réactivité aux évolutions du droit applicable aux prestations, il permettra d'assurer une meilleure équité de traitement sur l'ensemble du territoire et d'atteindre l'objectif de simplification des démarches pour les usagers, il contribuera également à l'amélioration de l'efficience du processus et un meilleur pilotage et suivi des dépenses de la de le système d'information commun est à la charge de la CNSA et le financement des briques national supplémentaire représente un coût supplémentaire pour la branche autonomie de 7 millions d'euros, dont les recettes sont annuellement votée par ce par cette mesure s'inscrit en cohérence avec la création d'un ici unique consacrée au versement de la pas et qui a été acté l'an dernier dans le cadre de la loi de financement de de la sécurité sociale pour 2022. Oui, donc c'est un avis favorable donc alors de de la part du rapporteur, puisque nous n'avons pas examiné en commission, puisque là, on est toujours dans la même logique, à la fois de modernisation et de simplification de la mesure en cohérence, a d'ailleurs avec la MDPH et rappelons que ça fait partie des outils fondamentaux pour pouvoir justement mettre en place une liste complète des besoins de l'offre et donc du pilotage et d'ailleurs, ça va être depuis très longtemps, donc voilà donc un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur, donc je mais aux voix l'amendement du gouvernement de 943 avec.

c'était un rapport qu'on a fait dans le cadre de la commission des finances, maintenant si nous sommes évidemment favorables au principe, je crois qu'il faudra être très attentif aux modalités de mise en oeuvre, parce que un système d'information, ça fonctionne aussi en lien Direct avec la façon dont les gens travaillent donc le ils sont organisés dans le service de MDPH pour monter les dossiers pour les examiner, il y a toute une organisation derrière tout ça, très complexe, elles sont différentes d'un département à l'autre, donc j'attire votre intention, Monsieur le Ministre, sur la nécessaire prudence et corrélation entre systèmes d'information et les façons de travailler, des départements, mais sur le fond, nous sommes favorables. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, le 1141 monsieur le Ministre. Si monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs. Je suis très heureux de vous présenter cet amendement puisqu'il est le le fruit d'un dialogue nourri avec les représentants des départements avec l'ADF, dont je salue le président François Sauvadet il s'agit par cette mesure qui vous est proposé de rehausser le plafond du concours de la CNSA qui permet à la CNSA de compenser aux départements une partie des coûts des revalorisations salariales. Des aides à domicile, dans une, dans un processus inverse à celui que vous avez décrit tout à l'heure et qui est d'ailleurs plutôt commun à l'ensemble des discussions que j'ai pu avoir depuis ma nomination avec avec les départements plutôt la dans un système de rallonge que de que de caisse qui serait pas dépenser, vous le savez la CNSA est historiquement aux côtés des départements et ces concours sont en forte. Tous depuis la création de la 5ème, branche de 3 milliards et demi en 2021, il est prévu qu'il dépasse les 5 4 milliards en 2026 soit une augmentation de plus de 50 % en 5 ans initialement limitée à la compensation de la paille de la PCH, ils se sont élargies à d'autres domaines, notamment le soutien au service d'aide à domicile, l'un de ces concours créé par l'article 47 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 permet d'accompagner les départements dans la mise en place des revalorisations actée par l'avenant 43 à la convention collective de la branche d'aide à domicile, en prévoyant un financement de l'État de 50 pour 100 de ces revalorisations, il vous est ici proposé d'ajuster ce soutien pour tenir compte de deux évolutions d'abord pour Tony, tenir compte de la décision prise à l'issue d'un travail de concertation que j'ai conduit avec les départements au sein du comité des financeurs, nous avons abouti à la décision d'augmenter la dose, heure à quatre euros dix ce qui représente un effort significatif pour la branche autonomie évaluée à 40 millions d'euros supplémentaires annuels cet effort je l'ai portée parce que je pense qu'il est indispensable de ne pas pénaliser mais au contraire de soutenir, d'inciter les départements qui font le choix de mener des politiques ambitieuses enfin en faveur du bien vieillir à domicile et donc de soutenir les opérateurs ensuite pour intégrer les coûts liés à l'extension des revalorisations salariales au service d'aide à domicile de la de la fonction publique territoriale, lesquels ont pris la forme d'un complément de traitement indiciaire acté au moment de la conférence des métiers de février 2022 cette extension entraîne des dépenses annuelles supplémentaires pour la branche de 21 millions d'euros, l'amendement proposant de relever le niveau du plafond de concours à 261 millions d'euros, soit 161 millions d'euros en plus c'est là encore le résultat d'un dialogue nourri avec l'ADF, qui a d'ailleurs été saluées par son président, tant pour sa méthode que pour son résultat et c'est surtout une mesure attendue par de nombreux départements et services d'accompagnement et d'aide à domicile, ces tarifs cet atterrissage symbolise, à mon sens la qualité du dialogue actuel entre le gouvernement et les collectivités. Merci, monsieur le Ministre, monsieur rapporteur. Monsieur le président, donc, très naturellement, ce sera l'avis favorable au titre en tant que qualité de rapporteur puisque nous n'avons pas vu cet amendement en commission et on a bien entendu que ça donc ça émane d'une concertation entre les départements et l'État, à l'occasion de la commission des financeurs du 27 octobre dernier on améliore de 61 millions d'euros, le transfert vers les départements. Mais simplement, au-delà de cette cette, je dirais de plus-values de la discussion, rappelons quand même qu'il y a encore un grand décalage entre les compensations entre l'État, les départements, donc on peut le saluer, mais à mon avis qu'un petit pas dans la négociation future, qui doit avoir entre l'État, les départements, surtout dans une perspective des d'évolution puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont sur la table, que ce soit en matière de PCH que soit en matière de bavardages, tout ça ce sont des coûts supplémentaires, et le principe général de le dire, c'est l'état qui décide les départements payent à un moment donné, nécessite des compensations à leur juste valeur, donc un avis favorable mais c'est qu'un c'est une ce n'est qu'un petit pas. Merci, monsieur le rapporteur, donc je vais aux voix l'amendement 1141 du gouvernement avec un avis favorable du rapporteur qui est pour. Qui est compte qui s'abstient-il être adopté l'amendement 274 Madame Mellow. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est nécessaire d'ouvrir les Epad vers l'extérieur et cet amendement est une suite logique, toutes les mesures qui ont été adoptés, l'accueil de jour permet au personne du territoire d'être accueillis souvent pour que les dents puissent souffler pour certaines personnes qui ont des troubles cognitifs et après avis du médecin coordinateur, ils pourront être admis à certaines activités du pôle d'activités de soins adaptés avec les pensionnaires de l'Epad, cela va dans le sens du maintien à domicile et de l'ouverture de l'Epad, sur le territoire, l'article D 312 du code de l'action sociale et des familles, précise simplement que l'Epasa accueille en priorité les résidents de cet établissement, rien ne s'oppose à l'heure alors à un accueil de jour, des personnes non résidente cet amendement propose d'accélérer le mouvement en créant une expérimentation. Monsieur le rapporteur. Mais c'est un avis favorable, donc, même si parfois ça se pratique sur le terrain, mais de le traduire par une exploitation sur 3 ans, donc voilà, avis favorable la. Monsieur le Ministre, Ministre, ce président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Votre amendement propose donc d'expérimenter pour une durée de 3 ans dans les pas à l'accueil de personne non résidente de l'Epad je partage évidemment votre double préoccupation de permettre une grande ouverture des Epad sur l'extérieur, mais aussi de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, notamment lorsqu'elle commence à développer des troubles du comportement, ces 2 objectifs s'inscrivent pleinement dans les politiques que nous conduisons visant à la fois accélérer le virage domiciliaires et de transformer les Epad il existe déjà un dispositif dédié à l'accompagnement de personnes âgées ayant des troubles du comportement et vivant à leur domicile, il s'agit des accueils de jour qui peuvent être autonome, ou bien adossés à des Epad ces accueils de jour ont un double objectif : répondre aux besoins de répit des aidants, des personnes âgées et proposer des activités tout à fait similaire à celle des pas Pour l'ensemble de ces raisons, la prise en charge que vous proposez me semble donc être satisfaite avec l'offre d'accueil de jour. Merci donc c'est un avis défavorable. Donc je mais aux voix l'amendement 274 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui. Pour qu'il est con. Qui s'abstient, il était adopté 4 amendements en discussion commune de 250 Madame Mellow. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ces dernières années, les engagements pris par l'État dans le cadre des revalorisations salariales, tels que le Ségur ou la hausse de l'inflation sont autant de sujets qui concernent l'ensemble des financeurs, tarification et de tarification du secteur social et médico-social dont la gouvernance est pluriel, ces mesures présentent des difficultés au niveau des collectivités territoriales, alors même que ces mesures ont été inscrites dans le droit positif, les gestionnaires des établissements du secteur de l'accompagnement social et médico-social ont ainsi besoin de gagner en visibilité sur les financements de l'ensemble des charges susceptibles d'impacter tant la masse salariale que les charges de gestion des établissements sociaux et médico-sociaux dans cette perspective, préalablement aux aux arbitrages relatifs au projet de loi de financement de la Sécurité sociale et au projet de loi de finances, il est utile de prévoir une conférence préalables réunissant l'ensemble des financeurs de l'action sociale et médico-sociale, cette conférence permettra de discuter de force façon collégiale des un engagement de l'État, des départements et des caisses de protection sociale afin de permettre aux gestionnaires du secteur, d'avoir une visibilité pluriannuelle des financements auxquels ils peuvent prétendre, et pour avoir l'objectif de l'État pour le financement effectif du grand âge elle précisera les modalités de mise en place des formations et de recrutement des 50000 employés prévus sur le quinquennat pour la prise en charge de l'autonomie. Le 330 Madame mascarade. Défendu merci le 90, la commission, monsieur le rapporteur. Merci président, alors c'est le même amendement simplement c'est la périodicité les autres abandons propose tous les ans, moi c'est tous les 2 ans. Je vais soutenir la l'amendement de la commission, mais, mais le plus important, il est pas là, il est surtout le message qui est porté à travers cette mise en place d'une commission pour quoi pour pourquoi proposé par la loi, c'est tout simplement parce que nous sommes dans l'attente d'une véritable loi sur l'autonomie et que, par défaut, hé bien on passe notre temps à voter PLFSS après PLFSS des mesures, brique par brique, sans vision globale, sans cohérence, on a même vu la voter la mise en place d'un outil de pilotage pour vous dire à quel point nous sommes en retard, donc voilà donc ces ces amendements surtout vocation à faire passer un message auprès du gouvernement ou je pense, quelles que soient les talents, les qualités des intervenants, quelles que soient les moyens financiers, si on n'a pas de vision globale, hé bien, on ne fait pas un bon une bonne politique, et donc je pense qu'il y a urgence, vous avez à travers vos interventions au moment de la discussion

l'accélération du vieillissement de la population quand même et concomitante du peu de progrès pour prévenir la perte d'autonomie, même on prend un grand retard sur la prévention de la perte de d'autonomie car si l'espérance de vie augmente l'espérance de vie en bonne santé ne connaît que des évolutions très modeste, à peine positives et de plus ça ne sont répartis très inégalement, nous y reviendrons pour pour un autre amendement selon les catégories professionnelles et les territoires pendant un temps, l'espérance de vie progressait plus dans l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, en fait une partie de l'espérance de vie gagnés et de plus en plus importante avec incapacité donc ces données doivent nous alarmer quant aux défis présents et à venir, le vieillissement de la population oblige à structurer rapidement ne drogue de soins aux conséquences, en lui conférant les moyens nécessaires, ça se cette cette conférence soit annuel parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard et préalablement aux arbitrages relatifs de façon annuelle du PLFSS et du PLF il semble utile de prévoir une conférence préalable réunissant l'ensemble des acteurs de l'action sociale et médico-sociale afin de permettre une discussion stratégique sur les orientations politiques et financières adopter en vue de céder des, des, des fils démographiques dans le code bien sûr d'une perspective pluriannuelle, donc c'était l'objet de cet amendement, qui avait d'ailleurs été je crois adopté par le Sénat en première lecture dans le cadre du Plfss 2022, sans toutefois passer le filtre de la navette qui sont pertinents, de lui donner une 2ème vie et moi je maintiens le caractère annuel, vu le retard que nous que nous prenons, d'année en année sur la prévention de la perte de tonus. Si cher collègue, Monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs, comme vous le savez j'ai lancé le 11 octobre dernier le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir 3 thématiques y seront abordés, celui de celles de l'adaptation de la société, celle de la question de la citoyenneté et du lien social et celle de la question de la revalorisation des métiers, la question d'une instance nationale de représentation des personnes âgées notamment fait partie des objets de la discussion, il me semble donc que votre amendement est un tout petit peu prématuré au regard de cette discussion. Merci, monsieur le Ministre, alors il y a demande de retrait Madame Mellow il est retiré au profit de celui de la commission 330 aussi madame salade. Donc 250 30 sont retirés le quatre-vingt-dix je fais voter sur l'amendement de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour, parce que cela varie pardon.

c'est bien trop tard, c'est bien avant les discussions qu'il aurait dû y avoir ça, quand vous pensez que vous avez mis des milliards d'euros pour la revalorisation des personnels dans le médico-social et que vous ne faites que des mécontents il y a quand même quelque chose qui va pas, si vous aviez organisé comme vous l'avez fait pour 61 millions d'euros, la discussion avec les les parties prenantes, et notamment les départements ben ça serait passé tout à fait de bonnes manières et vous n'auriez eu que des résultats positifs dans votre action, donc moi je ne crois pas qu'il arrive trop tôt, allons-y, c'est dès à présent qu'il faut, vers l'unité abonnement mettent les gens autour de la table. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté, donc il fait tomber le 933. Et nous poursuivons avec le 623 monsieur Fiole Oui, monsieur le Président, cet amendement réclame une évaluation du dispositif habitat inclusif afin d'avoir plus d'informations sur le recours réel à ce dispositif, un rapport de 2020 sur l'habitat inclusif a déjà dressé une liste de recommandations accueillie favorablement par l'ensemble des acteurs mais toutes leurs préconisations n'ont pas encore été appliqué, c'est notamment le cas de la majoration des aides individuelles au logement pour permettre aux habitants, aux ressources modestes de financer les espaces partagés cette évaluation permettrait de faire le point sur la mise en oeuvre des préconisations du rapport 2020 et d'avoir des retours sur les profils des bénéficiaires de l'habitat inclusif il permettrait ainsi d'identifier les besoins auxquels l'habitat inclusif n'est pas la réponse afin de formuler plus largement des propositions pour améliorer l'accès à tous à un logement adapté. Merci, monsieur le rapporteur. rapporteur. Demande de rapport dont sera un avis défavorable, et j'invite l'auteur de de cet amendement à lire attentivement le rapport pu tout Wolfromm qui dort, il y a plein d'éléments d'information. Donc c'est un avis défavorable

Oui, monsieur le président, donc, cet amendement prévoit la remise d'un rapport dressant un bilan de la refonte du modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile, prévu par la loi de financement de sécurité sociale 2022 valant l'opportunité d'exonérer d'après vous, c'est dur d'appels d'offres d'appels à projets les créations ou extensions des servir de tête et d'accompagnement à domicile dédié à l'habit. As inclusive, ça veut dire quoi, c'est que l'on va passer à une procédure d'appel d'offres, ce qui va faire que ça va figer les autorisations éventuellement accordées par les départements pour avoir des des Saad dédié à l'habitat inclusif et ça me paraît une bonne formule, pourquoi, parce que pour le plan du du personnel par exemple le personnel, il a des heures de de travail régulière, il sait qu'il est adapté, il y a un choix quand même qui est important et respecté également pour les personnes vivant dans l'habitat inclusif puisqu'elle fait peut faire appel, éventuellement un à un, ça extérieur et ça ne remet pas en cause l'avancée dans l'habitat inclusif, c'est la raison pour laquelle je pense que la procédure d'appel doivent être d'une complexité qui va pas aller dans le sens du développement de l'habitat inclusif, donc il vaut mieux le reporter comme on ne peut pas le faire, ça a pas été accepté au niveau des au niveau qui nous empêche de déposer des amendements, c'est sous forme d'un d'un d'un rapport, mais ce qui était important, c'est d'attirer votre attention pour qu'il y ait pas de retard par rapport à ces demandes d'autorisation pour les salles dédiées. Si monsieur le rapporteur. Sur les deux amendements demandant des rapports. l'a ouvert une possibilité, je dirais, d'avoir un outil adapté aux besoins mais par définition, on ira rajoute une contrainte administrative qui fait que de la souplesse qui était l'intention recrée la rigidité et donc je pense que c'est un point essentiel qui devrait être entendu dans la mise en place en matière de réglementation, voilà donc un avis défavorable sur les rapports mais très favorable sur le principe.

on diffère un peu sur sur les moyens d'abord sur la question du du rapport, la mesure qui vise à la réforme qui vise à prévoir la fusion des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, elle va entrer en vigueur, elle entre en vigueur et. Le décret définissant le cahier des charges de ces services devraient être pris au plus tard le 30 juin 2023, on l'a pas encore fait, là aussi pour pouvoir entamer une discussion avec les départements, donc la remise d'un rapport sur ce sujet serait un peu prématuré et quant à la question de la procédure d'appel à projets, je pense que c'est une une procédure utile, en tout cas, c'est ce que une partie des départements, m'ont dit pour permettent de sélectionner les projets correspondant aux besoins et aux priorités identifiées par les départements, notamment dans le cadre des schémas départementaux médico-sociaux, elle permet également de garantir une information suffisante à destination des acteurs de l'aide à domicile, ainsi que la transparence sur les critères de sélection des projets, l'objectif, c'est aussi de d'éviter la concentration de certains opérateurs sur ce type de sur ce type de, de, de dispositifs les personnes choisissant d'habiter dans le cadre d'un habitat inclusif peuvent recourir à des stades existants, comme toute personne âgée en situation ou en situation de handicap vivant à domicile, la spécialisation des Sade n'est donc pas une nécessité en terme d'accessibilité pour les personnes. Merci, c'est des avis défavorables merci Monsieur Savary. Oui, monsieur le Ministre, l'avantage des, des, des, de l'habitat inclusif, c'est que ça part du terrain. Je crois que, trop souvent, on est sur un schéma vertical, là, c'est quand même plus interactif, ça part du terrain, les départements peuvent définir un cahier des charges qui correspondrait aux projets qui sont proposés, émanant du terrain, c'est l'inverse de l'appel à projets qui définit tout et puis qui met en concurrence des gens qui demandent pas forcément que l'habitat inclusif se développe, se développe sur leur territoire, donc faut faire attentif à cela, et puis également, ça a l'avantage quand même d'éviter des déplacements et des kilomètres du personnel pendant ce temps là, il fait pas de son métier, on sait le coût que cela peut engendrer, donc je crois qu'il faut revoir entièrement ce dispositif surtout, surtout si on fusionne les ça dès l'Etihad parce qu'il y a pas besoin à ce moment-là, ça justifie d'autant plus, excusez-moi d'avoir des ça dédié à l'habitat inclusif parce qu'autant, elles ont besoin d'accompagnement ces personnes dans la vie quotidienne, qu'elles n'ont pas besoin forcément de structures de soins infirmiers, donc ça mérite une réflexion différente par rapport à ce qui a été menée jusqu'à présent et une prise de conscience des départements mais ça, il faut peut-être leur expliquer les choses de façon plus volontaire, me semble-t-il, merci. Merci monsieur le Président, c'est un amendement qui concerne les médecins qui existent exercent dans le secteur de la protection maternelle et infantile et de la santé sexuelle, nous sommes nombreux et nombreuses ici pointé l'intérêt de ce secteur en terme de prévention et donc ce qui est dans cet amendement, c'est pour que les médecins puissent bénéficier des des dispositions et de l'avancement dans le Ségur de la santé, c'est un sujet qu'on a évoqué il y a quelques jours ici, dans ce texte, la situation de la PMI très grave, il y a une diminution d'à peu près 24 % des effectifs qui est constatée entre 2010 et 2019 c'est l'étude de l'adresse, la détérioration du secteur de la santé périnatale est pointé aussi par le rapport de santé publique, France 2 septembre 2022, donc c'est une situation qui n'est pas normal et l'attractivité de ce métier doit être soutenue, donc c'est pour ça que nous demandons l'élargissement de la prime Ségur en complément traitement indiciaire pour les médecins territoriaux, dont ceux de la protection maternelle et infantile. Merci, monsieur le rapporteur. Alors c'est une demande de rapport donc sous le grand thème 10 oubliées du Ségur, vous savez que c'est un sujet récurrent depuis depuis la mise en place du Ségur, ça a été évoqué tout à l'heure, nous on était capable de mettre 3 milliards et demi sur la table sans réelle satisfaction dans l'ensemble des secteurs concernés, bon, quoiqu'il en soit, aujourd'hui, la, la demande de rapport concerne les médecins exerçant PMI et donc je voulais donner un avis défavorable, parce que sur cette demande de rapport mais pour pour gagner du temps par rapport au rapport, je propose qu'on pose la question au ministre directement sur le pourquoi est-ce que les médecins pays n'ont pas bénéficié de la prime Ségur. Merci, monsieur le Ministre, c'est le président, mesdames et messieurs les les sénateurs, madame la la sénatrice. Les médecins de PMI, à l'instar des médecins exerçant en établissements et services médico-sociaux ne sont pas concernés par cette mesure parce que il bénéficie depuis le premier avril 2022 d'un dispositif particulier de revalorisation correspondant à un montant brut de 517 euros, calculée sur la revalorisation moyenne des praticiens hospitaliers. Par ailleurs, de nombreux départements ont fait le choix de mettre en place, d'autres dispositifs de revalorisation des médecins de PMI et ne sont donc pas favorable à ce qu'un tel dispositif peut-être puissent être rendus obligatoire pour ces raisons je suis défavorable à votre avis. Merci donc je le mais au voile 417 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté de passons article 35 bis avec un amendement 345 Madame Bello. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on estime à 40000 le nombre d'enfants polyhandicapés ou ayant une paralysie cérébrale et accompagné par des établissements et services médicaux médico-sociaux en France, or les experts s'accordent à dire que la réadaptation et la rééducation de ses enfants, pour au moins la moitié d'entre eux, requiert une plus grande intensité de prise en charge, la création d'un parcours de rééducation et réadaptation coordonnées en ville, à destination des enfants polyhandicapés ou ayant une paralysie cérébrale vise à améliorer la prise en charge de ces patients sur le territoire français, de nombreux produits et services innovants en santé permettant d'optimiser la qualité de vie et le rétablissement de ses patients sont aujourd'hui développés par les industriels, mais les conditions d'accès au marché ne permettent pas toujours aux patients d'en bénéficier rapidement cette expérimentation de refonte des parcours de soins de rééducation et réadaptation doit être l'occasion de mettre à disposition des patients, les produits et solutions de santé les plus innovants et qui à l'heure actuelle, ne sont pas toujours accessible. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Ce, le président du point de vue de la commission, c'est un moment elle disait satisfait car je n'imagine pas que ces parcours de rééducation de l'adaption ne puissent pas bénéficier des produits les plus innovants, quoi qu'il en soit, la question est posée et donc, la Commission a conclu à une demande donc l'avis du gouvernement. Merci monsieur le ministre, monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice. l'intervention coordonnée de professionnels de santé conventionné ou non à vocation a assuré s'assurer de la prise en charge globale de ses enfants, et cela sans reste à charge pour les familles, le déploiement de ses compétences telles que prévues par le groupe de travail constitué d'experts constituera une réelle avancée pour ses enfants, cérébro-lésés et dit est polyhandicapé afin qu'ils puissent développer leur motricité et une fine et leur autonomie en outre un dispositif spécifique a été introduit il y a quelques années pour permettre maître la prise en charge de dispositifs médicaux présumé innovant en amont du droit commun justement pour pouvoir accélérer la mise à disposition patients de ces produits, en particulier sur le Champ de la compensation du handicap, donc vous dire que cette mesure est déjà en fait satisfaite par ce qu'on a déjà introduit dans la loi. Donc j'ai bien un avis défavorable à votre amendement Monsieur le président je devais retirer l'amendement mais nous serons vigilants parce que nous avions des eu des informations contraires, donc il faut être quand même très très vigilants sur le sujet. L'amendement 345 et donc je mets aux voix, l'article 35 bis qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté après cet article, l'amendement 610 monsieur Fiole R. Oui, monsieur le président, le texte de l'Assemblée nationale a introduit la création d'un parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, cette mesure ne répond toutefois que partiellement aux attentes des associations aussi cet amendement proposé par mon collègue Stéphane Artano vise à rappeler la nécessité de mieux accompagner l'ensemble des personnes avec paralysie cérébrale, à l'instar des centres de référence maladies rares, la création de Centres régionaux de compétences et de confiance pour la parasite cérébral permettrait de répondre au besoin de compétences des personnes avec paralysie cérébrale en assurant un suivi sans rupture de l'enfant à l'adulte vieillissant, deuxièmement de contribuer à l'éducation thérapeutique à l'information et la formation des acteurs du territoire, et enfin de développer la recherche appliquée. Monsieur le rapporteur. Un sujet intéressant mais comme si tu demandes de rapport, ce sera un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre même vie. Même avis parce que c'est prématuré. 2 avis défavorables, il est maintenu, le 611 je suis à la. Alors, malgré l'annonce d'une stratégie quinquennale d'évolution et de transformation de l'offre médico-social 2017, 2022, de nombreuses mesures prévues par le volet poly-handicap n'ont jamais été mise en oeuvre aussi cet amendement encore de notre collègue Artano demande un rapport d'évaluation du volet handicap de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre médico-social, ainsi que des propositions concrètes et budgété rappelle quand même que c'est une attente forte des associations qui réclament cette stratégie globale et. Merci, monsieur le rapporteur, c'est un sujet hein. Pourtant, mais que cette demande de rapport, un avis défavorable. Merci monsieur ce président, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur. Simplement, vous vous dire que, il y a eu un comité de pilotage le 8 novembre 2021 qui a permis de faire le point avec l'ensemble des parties concernées, en particulier les associations sur les réalisations acquises. à ce sujet, à cette occasion des axes de travail ont été identifiés sur lesquels les travaux, les travaux se poursuivent, tels que mieux documenter des besoins non pourvus à l'adéquation entre l'offre et les réponses attendues par les personnes et leurs familles, d'améliorer les pratiques professionnelles par l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques, publié par la HAS ou encore conforter la scolarisation des enfants pendant dix poly-handicapé ou poursuivre les travaux de recherche avec la cohorte de personnes polyhandicapés, là aussi, je pense que dans ce cadre, le rapport mais pas me paraît prématuré, donc je suis défavorable à votre amendement. Merci, il est retiré 600 osé retirer le six cent douze me suffit à l'air. La stratégie quinquennale d'évolution de l'offre médico-social 2017, 2022 comprenait un volet handicap psychique, il prévoyait notamment le développement de l'offre médico-sociale insuffisante dans de nombreux territoires, laissant des milliers de personnes sans solution d'hébergement ni d'accompagnement, ce volet n'a pas été mise en oeuvre aussi cet amendement invite le gouvernement à élaborer une réelle stratégie pour le handicap psychique avec une enveloppe budgétaire dédiée suffisante pour couvrir les attentes du public concerné. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur défavorable. Ceux de nouveau un avis défavorable sur ce rapport, mais de nouveau, je marque l'intérêt de la démarche, parce que là, nous avons vraiment pris du retard au regard des engagements qu'il a été pris par votre prédécesseur, voilà, donc je crois qu'il y a besoin de racheter et de et d'évoluer dans ce dans ce volet là sur l'évolution de l'offre pour ce type de handicap.

Alors, 75000 enfants naissent chaque année avec des troubles de neurodéveloppement l'ensemble de la communauté scientifique nationale et internationale recommande de mettre en place un programme de soins dès le repérage d'une anomalie de la trajectoire de développement, celui-ci doit pouvoir proposer sans attendent le diagnostic catégoriels parfois dès la grossesse de consultations spécialisées, la rééducation, un accompagnement éducatif co-construit avec les parents, ces interventions précoces multidisciplinaire en partenariat étroit avec les parents, permettent une amélioration de la trajectoire divers développementale et préviennent le sur-handicap permettant la construction d'une vie le la plus autonome possible donc dans cet objectif, cet amendement demande à nouveau un rapport sur l'accompagnement précoce des enfants naissant avec des troubles du neuro-développement afin d'évaluer les moyens en place et les besoins à couvrir. Merci, cher collègue, le 975 identique Monsieur Hassani il est défendu, c'est défendu, défendu merci, monsieur le rapporteur. Alors ce sera de nouveau un avis défavorable sur ces deux amendements que ces demandes de rapport, mais ça ne l'occasion quand même d'être le porte-parole des associations des des enfants qui sont concernés par les trous du neuro-développement. Qui s'clairement de ce Plfss et des moyens qui sont consacrés à la stratégie et l'évolution

particulière ce ce ce cet aspect-là, donc c'est à travers cette demande de rapport que nous pouvons relayer l'inquiétude tout simplement mais en tous les cas un avis défavorable sur la demande de rapport. C'est un sujet effectivement important et donc je je prends quand même quelques instants pour pour vous répondre, vous vous dire qu'il y a des mesures quand même dans le dans le PLFSS pour accompagner la mise en oeuvre de la stratégie autisme et troubles du neuro-développement qui arrive d'ailleurs à son terme et que nous sommes en train de, donc nous sommes avec une ambition là aussi renouveler parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est extrêmement important, je crois que, comme vous le soulignez le repérage de façon très précoce est nécessaire afin d'améliorer le développement de l'enfant et de prévenir le sur-handicap c'est pourquoi dans le cadre de la stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018, 2022, le gouvernement a fixé comme objectif la mise en place d'un parcours coordonné bilan et d'intervention précoce pour les enfants de 6 de 0 à 6 ans inclus afin d'accélérer l'accès à un diagnostic favoriser des interventions précoces sans l'attendre, et ainsi répondre aux problèmes d'errance de diagnostic et réduire les sur-handicap conformément aux recommandations de la HAS c'est dans ce but qu'ont été créés les plateformes de coordination et d'orientation des fameuses PCO les PC au zéro six ans sont en cours de déploiement sur le territoire et le dispositif était tendue depuis une instruction de 2021 aux enfants de 7 à 12 ans c'est PCO sont mobilisés, lorsque les médecins de première ligne suspecte un trouble du neuro-développement chez les, chez un enfant, les PC mettent en place alors des interventions adaptées et établissent le diagnostic, le bilan de la stratégie pour l'autisme au sein des TMD 2018, 2022 est en cours finalisation et donc j'ai le chiffre précis dans ce PLFSS on à 80 millions d'euros supplémentaires pour l'autisme et les troubles du neuro-développement or question de scolarisation de ces enfants tu ma féministe madame la salade. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous parle effectivement d'une amélioration de la prise en charge des troubles autistiques et du nord au développement, mais cette amélioration cette amélioration est-ce qu'elle devrait pas passer tout d'abord par la prévention, jusqu'aux années 2000 la prématurité, la grande prématurité n'a cessé de, d'améliorer sa prise en charge grâce à l'arrivée du surfacture de moyens qui ont permis au au pédiatre et animateur de, de, de, de réanimer correctement ses enfants, 2000, les années 2000, nous assistons à une dégradation de la prise en charge, à une baisse du nombre de pédiatres à une baisse du nombre d'internes en pédiatrie, ce qui fait que c'est souvent la la la la cause, la racine du mal, hein, soit pour ma grossesse, soit lors de l'accouchement, qui n'est pas prise en compte donc j'entends bien que vous mettez le paquet sur le, sur les conséquences quelquefois de cette mauvaise prise en compte de la périnatalité mais vraiment soyons logiques hein, on parle beaucoup de prévention, mettons le paquet sur cette période périnatale qui qui qui permettra de diminuer le nombre d'enfants polyhandicapés. Merci madame Cohen. Oui, je vais aller dans le prolongement de ce qui a été dit je, je, je pense que effectivement les mes collègues ont proposé plusieurs amendements qui du coup sont des demandes de rapport, puisque nous sommes, nous sommes bloqués par l'article 40 et en même temps c'est un cri d'alerte et d'alarme par rapport à la situation de ces enfants qui sont, qui sont nombreux et des familles qui sont parfois en déshérence, donc effectivement il y a une question de, de, de prévention, de diagnostic précoce et puis je je crois qu'il y a aussi une une une question très importante de rééducation de suivi, or j'attire votre attention, monsieur le le mini sur les fêtes sur le fait que notamment on est en manque de paramédicaux, je pense aux orthophonistes, alors vous allez dire je suis orthophoniste, donc je pense aux orthophonistes, mais il y a un manque cruel dans tous les établissements de cette, de cette profession et j'en profite pour dire qu'il faudrait réfléchir et desserrer le quota, c'est pas un numerus clausus, mais c'est un quota qui limite aussi beaucoup le nombre des orthophonistes et qui pénalise ses enfants en difficulté parce que quand on parle d'école inclusive quand on ne donne aucun moyen véritable pour accompagner ses enfants, on met ses enfants en difficulté et aussi l'ensemble des enfants de de donc il y a vraiment besoin de réfléchir de manière globale, en moyens financiers en moyens humains en formation aussi, c'est extrêmement important, et pas seulement se contenter de dire bon, voilà, ça y est on a réglé les choses de cette façon-là, quand j'ai commencé à exercer en orthophonie il y avait beaucoup de d'établissements spécialisés, le choix a été de les fermer, mais il ne faut pas se donner bonne conscience, comme ça, si on ferme des établissements ça nécessite que pour les pour l'école inclusive et pour l'accompagnement ça soit au contraire extrêmement renforcée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc voilà, je voulais profiter des amendements de mes collègues pour aussi intervenir sur ce. Oui, Madame Jouanno. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, on est là dans un passage, soit de propositions de de rapport ou de retrait, en tout cas, comment dirais-je d'avis défavorable de suppression et et je trouve que, en en réalité le nombre qui de rapports qui est proposé, nous interpelle parce qu'ils nous interpellent sur des sujets qui sont éminemment important, évidemment on ne peut pas intervenir parce qu'il y a l'article mais tous ces sujets font l'objet de, de, de, de, comment de questions qui nous interpelle tout au long de l'année, et notamment parce que nous avons l'occasion les uns les autres d'être nous-mêmes interpellé ou d'aller visiter des établissements qui qui nous interpellent sur ces sujets, je pense que c'est un manque d'informations souvent mais c'est aussi un manque de communication de la part du gouvernement, de nous dire où en sont les travaux et il faudrait certainement que vous puissiez intervenir un petit peu peu plus souvent en amont en en réalité est-ce que c'est pas des questions aussi écrite sur lesquels on n'a pas été enfin on on n'a pas eu de réponse je je crois qu'il faut s'interroger parce que là c'est ce n'est pas normal qu'on ait autant de demandes qui se suivent en fait ça, ça montre qu'il a quelque chose qui ne va pas, et il faut peut être en tout cas, notez la succession des sujets sur lesquels vous êtes interpellés, Monsieur le Ministre, pour pouvoir apporter des réponses complètes tout au long de l'année, merci. Merci, cher collègue, donc je mais se voit ces deux amendements identiques 613 975 avec 2 avis défavorables qui

d'article 40 qui s'est abattu un peu sur sur nos amendements et qu'on est obligé, oui, oui et que le le seul traitement qu'on a, c'est finalement de vous alerter et sur des sujets qui sont importants, pas simplement la prise en charge de ce handicap, mais même la prévention, on a vu un sur le prix natal le périnatale et vraiment, on attend des actions concrètes et d'être, a tenu informé.

Oui, monsieur le président, c'est de nouveau un amendement de d'une demande de rapport donc pour la suppression du d'un rapport concernant les relations salariales donc. Cap des Ségur des primes Ségur et désaccords Lafourcade au-delà de tout ça, je je fais relayé l'intervention de de de notre rapporteur général Madame Doineau sur le problème de l'information, voilà typiquement le sujet aujourd'hui, la plupart des des parlementaires si vous êtes pas spécialiste du sujet, où la plupart des acteurs sont complètement perdus concernant la revêt les hausses salariales

il y a le débat 10 oubliées du Ségur où on est interpellé partout, que ce soit le domaine du handicap du domaine de si on est interpellé partout parce que, malgré l'ensemble de ses efforts qui ont été faits, hé bien aujourd'hui il y a une liste de d'acteurs qui ne sont pas concernés Egon et au-delà du montant financier qui ont le scintillement de ne pas être reconnus dans leur métier, alors même que ce sont des métiers extrêmement difficile et qu'on passe notre temps à parler de valorisation et de revalorisation, c'est même pas un débat de, de, de, d'argent, c'est même si c'est important, c'est la reconnaissance de la nation, de l'importance de leur métier et je crois qu'aujourd'hui, il serait nécessaire d'avoir un tabou clair sur les interventions, un tableau clair ceux qui payent entre les départements et l'État, et surtout un tableau clair de ceux qui sont aujourd'hui écartés du dispositif de façon à ce que nous prenions conscience de la situation également des responsabilités du du du du gouvernement à travers tout ça, ça pourrait largement alimenté un rapport mais donc c'est une demande de suppression.

Oui alors, désolé monsieur le Ministre, moi ce tableau je le réclame depuis des mois et des mois et je n'ai jamais eu même pas actualiser donc j'attends avec impatience augmenter les salaires, c'était une très bonne chose, on était tous d'accord que la valorisation, la reconnaissance de ces métiers, passer par une revalorisation, ça on ne le remet pas en cause mais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est simplement la méthode que nous avons déploré alors tout à l'heure, vous avez annoncé une rallonge pour les aides à domicile, Monsieur le Ministre, moi j'aimerais entendre aussi qu'il y a une rallonge pour certains établissements, j'en viens évoquer la situation des établissements privés non lucratifs, moi j'ai été alertée par les dirigeants d'un Epad c'est les pâtes de Gacé, dans l'Orne pour ne pas le nommer, et avec la confirmation de la fédération du secteur, l'ensemble des établissements privés solidaire sont concernés par des carences de financement des différentes revalorisations annoncées par le gouvernement sur le financement du Ségura la revalorisation de 183 euros Net pour les personnels soignants des Epad : celui-ci est sous-calibrée depuis son entrée en vigueur en 2020 pour l'ensemble des établissements de la fédération du privé non lucratif, il manquerait 8 4 millions d'euros de financements en 2021, le décalage entre les financements et les besoins risquent d'être accrue en 2022 la FEHAP ayant été alertés d'une diminution des dotations de financement pour 2022 aussi Monsieur le Ministre, je vous exhorte à apporter une réponse forte et sans ambiguïté à ces établissements, en particulier parce que moi je sens un véritable découragement des professionnels mais aussi des bénévoles qui sont dans les conseils d'administration, en fait, là, ils y sont avec des Budgets vraiment difficile à tenir, je vous en conjure, il faut absolument les soutenir. et je crois qu'il est à jour dans l'annexe 5 c'est le point point puis le 2ème point quand je reprends tous ces débats récurrents régulier sur les Ségur sur les Lafourcade, etc, on parle de les 5 6 % peut-être d'un personnel qui ne seraient pas ou pas suffisamment revalorisé ou pas bien ou pas comme il faut, on oublie systématiquement les 95 % qui n'ont, qui ont été faits grâce au Ségur et qui n'avait pas été fait pendant les 20 à 30 ans auparavant et je me dis que, finalement, s'ils n'ont pas été fait pendant 30 ans, c'est peut être parce que ce qui est au pouvoir à cette époque-là avaient trop peur qu'on critique les 2 % restants merci. Merci, monsieur le Ministre.

que ces opérateurs et, ces établissements n'étaient pas, n'ait pas été compensé à l'Euro près sur les dépenses et les engagements qui ont été pris par l'état de de revalorisation pour ce qui concerne les départements, il y a des retards l'objectif est l'objet, en fait des de discussions que j'ai eu, dans le cas de du comité des financeurs à solder les comptes et à faire en sorte que, on puisse se dire : ben, maintenant il faut que les départements qui n'ont pas encore payé paye puisque l'État a effectivement répondu à à ses obligations et donc en plus de la compensation des 61 millions d'euros qu'on a inscrit tout à l'heure on a rajouté des crédits pour solder les obligations de l'État, suite à la conférence du 18 février dernier et donc une soulte de 14 millions d'euros sera versée et dispatché au département, selon la méthode qu'ils auront choisi d'ailleurs de calcul qu'ils auront choisi début 2023 et même chose pour les personnels des PMI, donc il il n'y a plus aucune raison aujourd'hui que ni l'État ni les départements ne respecte pas ses obligations, donc moi je veux bien que vous me vous me fassiez remonter directement les cas d'ailleurs chacun sur ces bancs, les cas que vous auriez en tête puisqu'on fait la chasse justement aux départements, aux ARS ou aux établissements

entraîner sur sur le terrain et c'est vraiment tout ce que je veux éviter à l'avenir, c'est pour ça que parmi là aussi, en plus de la réforme des concours de la CNSA on abordera dès le début d'année prochaine avec les départements, la question de la gouvernance globale, le pilotage de du secteur, notamment dans sa dimension masse salariale et pilotage conventionnelle, donc on prend le prétexte de l'accompagnement de la création du quatre conventionnel commun pour le secteur privé non lucratif pour mettre en place un cadre de gouvernance globale entre l'État et les les départements, les ARS pour pouvoir mieux piloter et faire en sorte qu'on ne reproduise pas ces difficultés demain et que par ailleurs on réponde aussi à la question de l'État prend des des décisions et sur des sur des compétences partagées et que les départements auraient a posteriori à financer sur sur leur parti, donc on a vraiment travaillé cette question de la gouvernance, qui à mon avis essentiel pour qu'on se retrouve pas dans cette situation et puis dernier point, on répond à l'urgence, encore une fois, enfin, l'objectif de l'État, et moi je l'ai passé à chacune des fédérations à chaque acteur que j'ai l'occasion de rencontrer, c'est de mettre en difficulté personne et a fortiori côté secteur privé non lucratif au secteur au secteur public vraiment qu'on soutienne tous ces opérateurs et donc il y a des mesures dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour répondre à la question de l'urgence liée à l'inflation, on a étendu le bouclier tarifaire sur les sur les Epad pour pouvoir faire face à l'augmentation des prix de l'énergie et on a donné des crédits supplémentaires aux ARS délégué des crédits supplémentaires aux ARS pour faire face à toutes les questions de d'augmentation liées aux approvisionnements divers et variés dans les dans les établissements scolaires. Si Monsieur le Ministre, dont je mais l'amendement 91 la Commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, donc, l'article est supprimé, article 35 inquiète le 92, monsieur le rapporteur. Oui, c'est une de nouveau, c'était un amendement de suppression d'une demande de rapport. Sagesse Monsieur le Ministre, monsieur le président, Mesdames et messieurs les. Sénateur avis divergent pour pour une fois on tient en fait à ce à ce rapport au regard du du du sujet qui est abordé, hein, qui est celui de, le, de l'évaluation des dispositifs d'appui de coordination, il me semble important de pouvoir bénéficier de de ce rapport, puisque l'unification des dispositifs d'appui à la coordination, ses 92

qui permettront ensuite de d'évaluer la nécessité ou pas. Suivre merci monsieur le Ministre, monsieur rapporteur. Oui, oui, contenant de cantonner la transmis j'ai retiré mon amendement, mais nous prenons acte dans le contrôle génétique de votre volonté, donc nous attendrons le rapport avec impatience pour une fois que l'État s'engage sur un rapport.

Alors, de nouveau, c'est une un amendement de suppression d'un rapport concernant la majoration de la PCH : je prends 20 secondes 30 secondes pour. Révoqué ce sujet essentiel, je vous rappelle que la PCH en dehors de ce qui concerne les aides humaine n'a pas été revalorisée depuis 2005 depuis sa création, donc vous imaginez le décalage dans le temps, au regard des coûts de l'inflation sur plusieurs années et il y a un vrai sujet va suer parce que la je vous rappelle de nous est à la charge en grande partie des départements et donc je comprends qu'on ne peut, on ne peut, par voie d'amendement, comme ça, augmenter la PCH, de nouveau d'avoir une vision globale, nous avions un premier outil qui date de 2005, nous avons ouvert la PCH aux troubles psychiques, l'année dernière de nouveau avec le sujet financier, je crois que ce point est essentiel pour qu'on puisse notamment répondre aux évolutions et aux demandes des personnes handicapées, mais dans le cadre d'une discussion commune État département sur le kiffait Dance quoi à travers cette évolution, donc leur demande donc de suppression du rapport, mais en tous les cas, un vrai sujet de à mon avis qui est nécessaire. Merci, Monsieur le Ministre. Ministre. Président, mesdames et messieurs les sénateurs à vie de sagesse du gouvernement, je voudrais simplement préciser que c'est un sujet qui va faire l'objet de discussions fournis dans le cadre de la préparation de la conférence nationale de du du handicap, qui aura lieu début 2023 tout cas ça fait partie des priorités qui ont été relevés que celle voilà de la compensation et des ressources de façon large des personnes en situation de handicap par le CNCPH. qui est contre. Qui s'abstient, il était adopté, donc il supprime l'article 35 sexy Yes 35 Sepp Thiès 94, monsieur le rapporteur. Demande également toujours une suppression de demandes de rapport sur un sujet analogue. Sagesse

moi je me rappelle il y a quelques années, ont touché 5 millions pour en dépenser 13 ça ne peut pas continuer comme ça, maintenant ça doit être pire que ça, c'est la raison pour laquelle, faut vraiment revoir cette dotation de départ qui est celle de 2005 revalorisé à l'Euro, je sais pas quoi selon la je ne sais plus quel critère mais qui ne correspond pas du tout à l'augmentation des dépenses pour les prestations nouvelles, donc c'est ça surtout parce que discuter, c'est bien beau, mais derrière faut sortir quand même, le carnet de chèques. Merci je mais aux voix l'amendement 94 avec un avis de sagesse du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté l'article 35 c'est pièce et supprimé après cet article, l'amendement 986 madame Meunier. Oui, rapidement, Monsieur le Président, puisque je connais le sort de cet amendement, mais tout cela pour dire, Monsieur le Ministre, que toutes ces discussions que nous avons aurait vraiment place dans une loi d'orientation du grand âge et de l'autonomie, plutôt que de voilà, voir des rapports se proposés se supprimer, c'est c'est bien dommageable, donc là ça concerne la part supplémentaire de CSG à la CNSA qui même si elle va dans le bon sens est largement insuffisante, vous avez l'évaluation les rapports, notamment le rapport de monsieur mais bien d'autres ont quantifié les besoins, nous les connaissons donc ce que nous demandons au gouvernement, hé ben, c'est d'avoir des garanties et en tout cas les intentions du gouvernement sur le niveau d'investissement dans le secteur médico-social, notamment pour tout ce qui est, recrutement de professionnels dans les EMS et dans au domicile qui ont fait l'objet de votre, de vos engagements récemment merci. Merci, monsieur le rapporteur. Donc un avis défavorable, entendu sur cet amendement, mais je soutiens en tous les cas, l'intervention de la Meunier. Merci, monsieur le Ministre. Avis défavorable du côté du gouvernement, même si je pense qu'il faut que nous puissions travailler pour actualiser affiner la trajectoire financière de la branche. Notamment au regard de toutes les discussions que nous avons ici dans le cadre de l'examen du projet, faire un peu la sécurité sociale que nous aurons également dans le cadre du CNR bien vieillir pour déboucher sur ceux qui seront des mesures éventuellement législatives d'ici à l'année prochaine. qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 36, une prise de parole du rapporteur Monsieur Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, je veux pas reprendre les arguments qui ont été exposés lors de la discussion générale, mais quelques mots quand même pour cet pour cet article 36 qui inaugure les dispositions du Plfss concernant la branche familiale, la branche famille, comme annoncé, la commission a a soutenu l'évolution du complément de libre choix du mode de garde qui devait réduire le reste à charge pour les familles aux revenus les plus précaires, permettez-moi toutefois de réitérer les doutes, je dis le doute plutôt que griefs qui laisse un goût d'inachevé à cette réforme, je crois d'ailleurs que ces doutes sont largement partagé dans cet hémicycle en voir les nombreux amendements déposés initialement mais recevables financièrement sur ce sujet : d'abord la mise en oeuvre de la réforme induit des perdants sur lesquels nous avons peu d'informations, or le mécanisme temporaire de compensation est doublement plafonnée, d'une part par une condition de ressources et d'autre part, il est réservé aux familles, recourant à un nombre minimal d'heures de garde ensuite l'ambition de la réforme que vous nous proposez monsieur le ministre aurait pu être rehaussé l'article 36 permet aux familles monoparentales, de recevoir le CMG emplois Directs jusqu'au 12 ans de leur enfant, contre 6 ans pour le droit commun, c'est bien, mais cette possibilité aurait pu être étendu à d'autres familles en situation de fragilité, rendant difficile la conciliation de leur mode de vie familiale et professionnelle, je pense par exemple au parent bénéficiaire de l'adulte deux lacs location adulte handicapé de la prestation de compensation du handicap ou enfin de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé alors j'ajoute que, vous savez, j'avais un maître, j'ai un maître André Diligent qui a été sénateur ici assez longtemps qu'il était maire de Roubaix qui disait qu'il y avait 3 choses importantes : c'était le calendrier, le calendrier et le calendrier et donc regretter que cette réforme soit seulement en vigueur dans trois ans, je vous remercie, merci Madame Cohen. Si Monsieur le Président, l'article 36. Forme le complément de libre choix du mode de garde et prévoit notamment l'extension de la prestation jusqu'au 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales et prévoit un meilleur partage la prestation en cas de gale garde alternée de l'enfant, comme ça a été rappelé l'augmentation du complément de libre choix du mode de garde favorisent les solutions de garde par emplois Directs d'une assistante maternelle ou d'une garde à domicile, si cette mesure peut améliorer la situation des familles nous voulons relayé ici les craintes des associations familiales sur l'effort politique qui devrait porter prioritairement sur les établissements d'accueil du jeune enfant dont l'offre en terme de place est structurellement insuffisante pour répondre aux besoins des familles, je rappelle que le déficit de places de crèches et haltes-garderies est estimé aux alentours de 250000 places alors que 60 % des enfants sont gardés chez une assistante maternelle, en raison aussi de ce manque de de places de crèche, la revalorisation du complément de libre choix va envoyer un signal positif aux familles mais négatifs aux collectivités, ce progrès pour les familles ne doit pas masquer en réalité, Monsieur le Ministre votre timidité pour ne pas dire votre renoncement à tenir vos engagements par rapport à l'ouverture de places de crèches, selon l'Union des familles laïques, le signal envoyé aux collectivités qui subissent déjà l'augmentation des prix de des prix de l'énergie et de renoncer à ouvrir de nouvelles places de crèches donc soyez attentifs à ça, monsieur le ministre est d'autant que vous prévoyez le transfert de 2 milliards d'euros de la branche famille à la branche assurance maladie sur les indemnités parentales et même si le Sénat s'y avec le 49 3 que vous dégainez assez facilement à l'Assemblée nationale, je crains que notre refus collectif soit balayé. Merci, cher collègue, l'amendement 96 rédactionnel, monsieur le rapporteur. le premier amendement est un amendement rédactionnel effectivement. Miss favorable, favorable, il y a pas d'opposition, l'abstention, il est adopté le 96 nous passons au 95 avec un sous-amendement de 138, monsieur le rapporteur. Alors il s'agit donc d'un amendement qui concerne les assistantes maternelles qui font face à une multiplication d'impayés de leur rémunération, c'est un sujet que nous avons beaucoup entendues lors des auditions la CNAF nous a d'ailleurs confirmé avoir connaissance de cette recrudescence et ses assistantes maternelles se trouve en difficulté pour obtenir gain de cause, lorsque la famille n'adhère pas l'intermédiation par page, j'emploie le le complément de libre choix du mode de garde continue dans ce cas être versée aux familles et, donc, cet amendement vise à suspendre sans délai le versement du CMG au foyer qui ne se quittent pas du salaire de l'assistante maternelle ou de la personne employée pour un, un, une garde d'enfant à domicile, ces dernières ont alors la possibilité de signaler cette situation à la CAF ou à la plateforme Pajemploi il s'agit d'une première avancée que la commission propose mais ces situations d'impayés sont inacceptables et elles ne trouveront des résolutions rapides que c'est le gouvernement et la CAF prenne les dispositions nécessaires pour accompagner les professionnels de la petite enfance, je vous remercie. Oui, donc il est dans la prolongation de de l'amendement de du rapporteur quant à ses à payer quand même, je souhaitais rappeler la rémunération des assistants maternels qui s'élevaient en moyenne selon l'adresse alors on n'a que 2014, je ne comprends pas qu'on ait pas de données plus récentes à 1108 euros Net année où 58 % des assistants maternels qui travaillaient à temps complet percevaient moins de 1250 euros Net par mois,

l'amendement bienvenue du rapporteur Olivier Henno, vise à tenir compte de ces sujets de ces situations où, effectivement, le salaire n'est pas versée, mais où, paradoxalement, enfin la CNAF continue de verser le CMG aux parents, aux parents en suspendant donc le versement de du CMG, je propose d'aller plus loin par ce sous-amendement car depuis plusieurs années sa famille en place ce service page emploie plus qui permet de confier à l'organisme public l'intégralité du processus de rémunération de du salarié en tenant compte des prestations familiales auxquelles l'employeur peut avoir droit en 2021, le dispositif concernait environ 400000 assistantes maternelles si l'intérêt de ce service n'est plus à démontrer, en terme de facilitations administratives, notamment pour le parent employeur, il permet aussi de sécuriser et et de rendre régulier le paiement du salaire de 100 maternels, donc cet amendement vise à renforcer les dispositions de l'amendement du rapporteur via l'obligation pour l'employeur ayant été visé

Alors je vais pas redévelopper l'objet de l'amendement, je pense qu'il a été explicitée de façon suffisamment précise mais dire que ce dispositif nous a semblé intéressant et donc parce que pas emploie est une garantie supplémentaire que la rémunération du professionnel sera versée l'Urssaf déduit alors le montant CMG de la rémunération et prélève directement, le reste à charge sur le compte bancaire bancaire de la famille, employeurs et donc pour cette raison, nous émettons un avis favorable, je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de revenir de façon générale sur cette réforme du CMG, qui est une réforme extrêmement ambitieuse, vous voyez le gouvernement investit pour accompagner les familles dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 1 milliard 600 millions d'euros de mesures dont cette réforme du complément mode de garde qui est la première brique du service public de la petite enfance, qui est une promesse du président de la République de créer d'ici à 2030 200 places en crèche comme auprès d'assistante maternelle, puisque je vous le rappelle aujourd'hui, 200000 places. D'accord. Puisque je vous le rappelle, j'ai pris avec des chiffres, je vous le rappelle. Aujourd'hui 60 des places sont portés par les assistantes maternelles auront c'est que on va en avoir besoin de beaucoup demain si on veut atteindre ses objectifs, en particulier au regard de in attractivité du métier, mais également d'une courbe démographique qui nous est extrêmement défavorable, c'est pour ça que ce complément mode de garde vise d'abord à rendre le reste à charge pour les familles équivalent qu'on mette son enfant en crèche ou qu'on mette son enfant chez une assistante maternelle, ce qui permet d'ailleurs un accès pour les familles les plus modestes, ce mode d'accueil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a décidé cette mesure d'extension pour les enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, on assume un choix clairement social pour accompagner les familles les plus en difficulté, les plus modestes, j'entends monsieur le rapporteur, vos questionnements sur le dispositif de transport de de transition sur l'impact de la réforme sur les ménages, a fait, on a fait des des projections, le timing, le temps de mise en oeuvre de la réforme va nous permettre de conduire les concertations et les les études nécessaires pour assurer un impact le plus minime minime possible pour encore une fois les familles modestes et de classe moyenne, il est vrai qu'on a fait le choix d'être un peu moins protecteur vis-à-vis des familles plus aisées et en particulier celles qui bénéficiaient, on va dire de d'aide et d'un complément mode de garde dans les modes de garde individuelle qui était supérieur à celui qu'on pouvait trouver dans les crèches concernant la rémunération des des assistantes maternelles, les chiffres que nous avons, nous, plus récent, qui date de 2021 et notamment ceux qui sont présentés par l'UNSA ce matin suite à leurs études font état d'un salaire moyen pour les assistants maternels de 1495 euros Net par mois, donc voilà et donc il y en a qui gagnent un peu plus, il y en a qui gagnent moins, mais voilà, le salaire moyen et demi quatre cent j'ai réuni d'ailleurs, c'est les assistantes maternelles, pas plus tard que cette semaine en début de semaine pour évoquer avec elle, l'avenir de de leur profession et notamment ces ces questions et je peux vous dire qu'elles sont extrêmement satisfaite de fait de cette réforme qu'elles attendaient depuis extrêmement longtemps concernant l'amendement du du rapporteur votre amendement met en lumière la situation de parents employeurs qui ne respectent pas les termes du contrat de travail avec le salarié, assurant la garde de leur enfant, en d'autres termes, de parents qui ne reste. Affecte pas le code du travail qui s'impose à tous les employeurs, il s'agit là de situation indigne contre lesquels nous devons bien sûr lutter, je souhaite d'abord rappeler qu'en l'état actuel de la réglementation, l'absence de dépenses effectives par le par employeur n'ouvre heureusement pas droit au versement de la prestation, la déclaration d'un salaire versé dans le dispositif Pajemploi sans versement effectif du salaire est en effet constitutif d'une fraude et donne lieu à récupération des sommes indûment envers versée par les caisses de Sécurité sociale, je souhaite également souligner qu'ayant été informés à plusieurs reprises ces dernières semaines de ces situations d'un d'un payé, j'ai échangé avec les représentants associatifs et syndicaux, des assistants maternels, afin notamment de recueillir leur point de vue sur cette question, il ressort de ces échanges dont je tiens un compte rendu, à votre disposition ainsi qu'un courrier qui m'a été adressée par FGT à FO, que la plupart de ses représentants, représentants, estime que le dispositif que vous proposez ne se ne suffirait pas à répondre à la problématique qui est la leur, en ce qui est sans effet sur la situation de l'assistant maternel, la suspension du versement du CMG ne permettant aucunement de rétablir le versement du salaire ni de rechercher les sommes dues au titre du travail réalisé les représentants des assistants maternels moins cette occasion confirmé plutôt leurs voeux pour un mécanisme de garantie des salaires, appelé à être discuté par exemple dans le cadre du comité de filière, petite enfance, qui rassemble employé employeur et de manière plus générale, toutes les parties prenantes du secteur j'ai par conséquent demandé à sa présidente, Madame Élisabeth laitier de prioriser le traitement de ce problème en vue qu'une réponse opérationnelle y soient apportées dans l'année pour ces raisons je suis défavorable à vos amendements. Merci, monsieur le Ministre, donc je mais aux voix l'amendement le sous-amendement 938 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté et je mais aux voix l'amendement 95 de la commission 6 sous-amendé avec un avis défavorable du gouvernement qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient il être adopté l'amendement 97, monsieur le rapporteur. pour le bénéfice du CMG donc ce plafond a été créé par la LFSS de dès 2014 et il est plafonné à 10 euros depuis maintenant 2016 et ça pose évidemment des problèmes d'actualisation, compte tenu du contexte économique, compte tenu de l'inflation également et donc, cet amendement vise à remédier à cette situation, obligeant le gouvernement a fixé chaque année ce plafond après avis du Haut Conseil de la famille de l'enfance et de la je vous remercie. monsieur le le président, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le. Le rapporteur. Et donc vous proposer que le gouvernement fixe chaque année après avis du HCA le plafond limitant le tarif horaire des micro-crèches afin d'améliorer l'efficience de la politique de création de places de crèches, je partage évidemment les la nécessité de permettre le développement et la solvabilisation de structures d'accueil du jeune enfant, toutefois, il convient de rappeler en 1er lieu que le CFE-a dans son décret constitutif ne rend des avis que sur les projets de nature législative afin d'apporter aux acteurs publics une expertise prospectives et stratégiques complémentaires de par son positionnement et sa composition étendre ses missions à une compétence d'avis isolé sur un Quantum financée de nature réglementaire me semblerait peu cohérent, par ailleurs, l'objectif du plafond de 10 euros et de concilier l'accessibilité financière au micro-crèche pour l'ensemble des familles et non les seules familles les plus aisées avec la soutenabilité du modèle économique de ces acteurs de l'accueil du jeune enfant le con où le gouvernement a déjà eu l'occasion d'informer les gestionnaires de micro-crèche qu'une discussion sur la soutenabilité économique de leur modèle ne pourrait être, à mon sens s'engager qu'une fois communiquer des informations suffisamment précises sur le niveau de leur coût de revient ce don, enfin, nous n'avons pas communication à ce stade seyant donc ces éléments n'ayant pas encore été transmis j'émets un avis défavorable à cet amendement. Merci, monsieur le Ministre, donc je baise aux voix l'amendement 97 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté je mais au voir l'article 36 ce qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Après cet article, 2 amendements discussion commune de 232 Madame Procaccia. Oui, merci Monsieur le Président, l'article 36 sur la CMG, nous semble-t-il, ne concerne pas les services prestataires de garde d'enfants ou l'intervenant et directement employé par un service et qui a un maillon essentiel de l'offre pour permettre aux parents d'accéder une solution de garde, c'est la raison de cet amendement et de cette demande de rapport, sauf si vous nous expliquez que ses services sont bien inclus. discussion commune oui le 739. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le projet de loi prévoit des le bénéfice du CMG aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, car les dispositifs d'aide à la garde sont limitées, alors même que les enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle reste important cette problématique se pose également pour les parents d'enfants en situation de handicap de façon d'autant plus prégnante que nombre de ses enfants ne bénéficient pas d'une scolarité à temps plein, alors que ceux qui sont scolarisés dans une unité d'enseignement médico-social ne bénéficient pas d'activités périscolaires après 16 heures 30 et que l'accès au centre de loisirs et de vacances ne sont pas toujours une réponse facile à mobiliser, faciliter l'accès des familles dont les enfants situé à sont en situation de handicap ayant des enfants âgés entre 6 et 12 ans, en est à un mode de garde formel constitue là aussi un enjeu majeur en terme de soutien de la conciliation de leurs différents temps de vie d'accès et de maintien dans l'emploi et donc de levier de sortir de la pauvreté mais aussi faut se le dire, chers collègues de répit pour les familles par cet amendement, nous tenons donc à alerter sur la nécessité de mieux prendre en compte les besoins des enfants et des familles dont un enfant est en situation de handicap, même si on ne se fait pas d'illusions sur la sur le vote pour ce rapport, merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président, Monsieur le ministre, on a compris depuis ce matin, qu'il est arrivé qu'on refuse des rapports sans marquer un désintérêt pour la question évoquée, donc ce sera un avis défavorable je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le le président, mesdames et messieurs les les sénateurs avis défavorable sur le premier amendement puisqu'il propose un rapport pour. S'agissant de mesures qui n'entreront pas en vigueur avant 2025 et donc un rapport pour 2024 ce qui semble un tout petit peu prématuré et que, par ailleurs, au regard de l'ampleur de de la réforme, je préférerais qu'on puisse avoir le temps de la mettre en oeuvre avant d'en on envisager l'extension du le le l'amendement pardon du sénateur Iacovelli vous proposez donc que le Gouvernement remette, là aussi, avant le 1er janvier 2024 un rapport dressant le bilan des réformes du CMG qui vous sont proposés, n'arrive qu'ils ne seront mises en oeuvre, pas avant 2025. En ce qui concerne l'extension aux familles avec enfants en situation de handicap du CMG 6 12 ans je tiens à vous indiquer qu'un certain nombre de dispositifs existent déjà parce que c'est un vrai sujet, comme vous l'avez souligné pour les modes de garde avant six ans ces familles bénéficient d'une majoration des montants du plafond du CMG et d'une minoration du taux d'effort supporté en cas d'accueil en crèches par ailleurs elles peuvent bénéficier d'aides de la branche famille, y compris au-delà de 6 ans de l'enfant, dédié aux surcoûts induits par ces situations, je pense par exemple à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou encore à l'indemnisation des congés pris pour s'occuper de l'enfant, les parents en situation les parents en situation de handicap bénéficient eux aussi de dispositifs spécifiques, je pense en particulier à la PCH parentalité qui permet de bénéficier d'une aide humaine et d'acheter du matériel adapté. Pour pouvoir s'occuper de son enfant, je pense également au crédit d'impôt, service à la personne dont le plafond de dépenses éligibles à augmenté pour certaines personnes invalides à la déduction forfaitaire de cotisations patronales ou encore à l'aide au recours à un prestataire pour des personnes handicapées ou l'évolution de ces dispositifs déjà nombreux me semble relever des discussions qui auront cours lors du prochain conseil national la prochaine pardon conférence nationale du handicap en début d'année prochaine, pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement ou à défaut je ne pourrait qu'être défavorable.

Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est un amendement qui est un peu plus qu'un amendement rédactionnel qui ce qu'il prévoit, comme l'année dernière un alignement pérenne des conditions d'accès d'accès des fonctionnaires aux congés sur celle prévues dans le code du travail, je vous remercie, monsieur le monsieur Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur, votre amendement donc vise à aligner totalement sur les salariés, les conditions d'accès des fonctionnaires au congé de présence parentale, c'est l'harmonisation entre secteurs public et privé public et privé est, évidemment, à rechercher, et c'est ce que nous faisons avec cet article, il apparaît nécessaire de l'articuler avec les spécificités de la fonction publique, par exemple, contrairement au secteur privé, le congé de présence parentale ne peut être fractionné par demi-journée, dans la fonction publique au regard de la règle transversale du 30ème indivisible, par ailleurs, en effectuant un renvoi au code du travail, votre amendement entrave l'objectif de lisibilité du droit qui était recherché par le nouveau code général de la fonction publique, celui-ci réunit l'ensemble, pardon, l'ensemble des dispositifs applicable aux fonctionnaires dans le même corpus juridique et qui serait complexifié par un tel renvoie pour ces raisons je suis défavorable à votre amendement. Merci monsieur le ministre. Donc je mais aux voix l'amendement 98 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Président. Il est adopté. Madame la présidente, il y avait un problème. et un problème d'affichage, on veut aller vite, mais pas si vite que ça. Donc, en réalité, donc l'amendement 98 a été adopté et donc l'article 36 bis, je le mettre aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté même vote pour le trente Sister même vote il est adopté au 36 squatter un amendement 99 de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, il s'agit de de la suppression de de cet article, puisque cet article ce bonne se borne monsieur bonne à modifier le caractère explicite de l'accord du service du contrôle médical sur la demande de renouvellement d'un congé de proche aidant, il n'a ainsi aucune incidence sur les comptes de la Sécurité sociale et paraît il recevables au regard du domaine des lois de financement de la Sécurité sociale, par conséquent, cet amendement propose la suppression de cet article, Merci, monsieur le Ministre, c'est le président, mesdames et messieurs les sénateurs Monsieur. Le le rapporteur et nous donc vous proposez de supprimer cet article créé à l'initiative du rapporteur Paul Christophe à l'Assemblée nationale et qui prévoit la suppression de la condition d'accord explicite pour le renouvellement exceptionnel de lâche comme vous le savez, la possibilité de renouveler les droits à l'AFPA a été ouverte l'année dernière par une loi portée par Paul Christophe, cette proposition avait été largement soutenue dans cet hémicycle, et je crois d'ailleurs que vous en avez souligné l'importance le nouveau dispositif vise à améliorer la situation des familles qui accompagnent un enfant dont la dégradation de l'état de santé résultant d'une pathologie telle qu'un cancer pédiatrique, par exemple, d'un handicap ou d'un accident particulièrement grave se poursuit au-delà de 310 jours, or l'accord explicite du service de contrôle médical pour renouveler la durée de perception de l'AJPP. C'est identifié dans la pratique, comme une lourdeur administrative pour ces familles fragilisées qui font déjà face à une situation critique, de nombreuses familles associations ont fait remonter ce point point quant est confrontée à la maladie de son enfant, le rôle des pouvoirs publics et de faire le maximum pour l'accompagner dans cette épreuve, épreuve, notamment en facilitant ses démarches pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à son enfant l'évolution que propose cet article et donc d'une importance cruciale pour les familles qui voit l'échéance du renouvellement s'approcher, parallèlement à la maladie de leur enfant, s'agissant de la place en loi de financement de la Sécurité sociale de cette mesure, je ne partage pas tout à fait votre analyse, dans la mesure où cet amendement vise clairement à accroître le recours à l'AJPP, cette prestation, comme vous le savez est entièrement financé par la branche famille, je suis donc défavorable à votre amendement. Merci, monsieur le Ministre, dont je mets aux voix cet amendement 98 de suppression de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement de la commission vous propose de supprimer cet article 37 qui rend obligatoire le versement par l'employeur au salarié d'une somme au moins égale aux indemnités journalières du pour les congés ou maternité d'adoption et de paternité, l'employeur serait ensuite sub-Roger dans des droits des assurés de percevoir des indemnités cette à cette option peut être utile pour les bénéficiaires des accords de branches peuvent le prévoir où les entreprises peuvent choisir librement de mettre en place ce circuit financier cependant une telle obligation légale semble disproportionnée, elle fait peser des coûts de trésorerie aux employeurs sans distinction des entreprises, les TPE et les PME ou les entreprises à la trésorerie sous tension seraient concernés, de plus, cet article ne paraît pas avoir d'incidence directe sur les comptes de la Sécurité sociale et donc, nous vous proposons de supprimer cet article, j'ajoute que pour les quatre amendements qui suivent, c'est bien sûr un avis favorable.

Défendu, c'est le même, le 675 défendu aussi monsieur mouiller le 972 n'est pas défendu, il tombe. Donc sur ces quatre amendements identiques. Le ministre, monsieur le président, Mesdames et messieurs les. Les sénateurs, vous le savez, l'accueil d'un enfant dans une famille et il est un moment parfois sensible et délicat, c'est pourquoi il nous faut garantir les ressources du foyer à ce moment-là de de la vie. C'est d'autant plus le cas quand nous encourageons et c'est bien la volonté du gouvernement la prise par les parents de la totalité de leurs congés maternité ou paternité, donc je rappelle que la durée a été doublé à 28 jours depuis le 1er juillet 2021, le calcul de l'indemnité journalière versées lors d'un congé maternité est proportionnel aux revenus des salaires hors les éléments de paye sont parfois transmis tardivement par les employeurs aux caisses primaires d'assurance maladie, ce retard explique les longs délais de versement aux assurés, en effet, une fois que l'assurance maladie disposent des éléments de salaire, elle ne met que 7 jours à verser des indemnités journalières, c'est pour répondre à ces difficultés que le gouvernement vous propose cet article 37 37 gouvernement a conscience des difficultés de trésorerie dont certaines entreprises pourraient faire état, c'est pourquoi la mesure prévoit également une garantie. Paiement rapide des employeurs dans un délai qui serait déterminé par voie réglementaire, en contrepartie de ce maintien de salaire et pour limiter l'impact en trésorerie, la mesure impose un délai de remboursement par ailleurs la mesure laisse le choix à l'employeur de choisir le levier de remboursement en fonction de l'organisation interne de son entreprise, ainsi l'employeur qui ne souhaite pas être sub-Roger peut en échange du maintien de salaire exercer une retenue sur salaire, au retour de congé de son salarié, l'employeur pourra donc choisir de se faire rembourser l'avance de salaire, soit par subrogation soit par une retenue sur salaire, il ne s'agit pas un transfert de missions de la sécurité sociale, aux entreprises, l'assurance maladie continuera de calculer l'indemnité journalière afin de rembourser à bon droit, le montant avancé par l'employeur, enfin, le gouvernement a prévu une mise en oeuvre échelonner dans le temps afin de les laisser notamment, afin de laisser notamment aux petites et moyennes entreprises, le temps de s'approprier le dispositif des concertations avec les partenaires sociaux ont relié au 1er semestre 2023 afin de partager le contenu du décret qui doit définir le périmètre des employeurs concernés le rythme d'entrée en vigueur et les modalités de mise en oeuvre le retard d'indemnisation ne doit pas être un frein au projet de fonder une famille, le maintien d'une rémunération au moins équivalente au montant des indemnités journalières permet d'y remédier, enfin en ce qui concerne la remarque sur la place d'une telle mesure dans la loi de financement de la Sécurité sociale, je souhaite également indiqué que la garantie de paiement et la réduction des délais de paiement de l'employeur ce Breger ont bien un effet sur la trésorerie des organismes de Sécurité sociale, l'augmentation induite du taux de recours au congé paternité aura par ailleurs un impact en dépense au regard de l'impact sur les familles de cette mesure, vous comprendrez que le gouvernement tient particulièrement au maintien de cet article 37. Merci monsieur le ministre, monsieur mouillé. Oui, monsieur le président, rapide, d'abord pour et vous. Puis aussi la difficulté pour les petites entreprises, des démarches administratives, c'est-à-dire de nouveau au-delà du de la trésorerie, on rajoute ou petites entreprises finalement une mission qui a été porté par la sécurité sociale, donc je suis pas sûr bon signe, et de nouveau, moi je reviens sur la méthode, la méthode de ce gouvernement qui a pas beaucoup changé, parce qu'on vote un texte et après on va faire les concertations avec les entreprises, donc, de nouveau, je pense qu'on aurait préalablement dû discuter avec le bras entend des TPE, des PME avant d'élaborer les sujets là on va voter le texte et le décret les décrivent les allez négocier dans les premiers prochain semestre, je trouve que la moto encore douteuse. Merci, cher collègue, donc je mais on voit. Les amendements 100 242 351 675 identique avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés et donc l'article 37 et supprimé, nous passons à l'amendement 737 avec monsieur Oui, Monsieur le Président, cet amendement est un amendement d'appel et qui propose d'engager une réflexion visant à empêcher qu'un couple avec enfants dont l'un des parents est en situation d'invalidité, de se voir retirer le droit à l'allocation de base de la Paje sous prétexte qu'une pension d'invalidité des constitue pas un revenu d'activité avec un enfant, le plafond de ressources 2020 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 retenue pour le calcul de l'allocation de base à taux plein et de 27219 euros pour un couple avec un un seul revenu d'activité et de 35960 et 11 euros pour un couple avec deux revenus d'activité, par exemple un couple dont l'un des dans l'un des parents est en situation d'invalidité partielle et qui perçoit encore un revenu d'activité peut percevoir cette allocation, pour peu que les ressources Net imposables du foyer ne dépasse pas le plafond pour un couple avec deux revenus d'activité, en revanche en qu'un d'invalidité totale d'un des 2 parents, bien que la pension d'invalidité soit comptabilisés parmi les ressources Net imposable, elle ne constitue pas un revenu d'activité en ce sens, le plafond qui s'applique pour le calcul de l'allocation est celui d'un couple avec un seul revenu d'activités, c'est-à-dire 27219 euros ainsi malgré des ressources nettes imposables presque inchangé, un couple où l'un des 2 individus devient invalide peut se voir retirer le droit à l'allocation de base de la Paje sous prétexte qu'une pension d'invalidité ne constitue pas un revenu d'activité ainsi je vous propose d'engager une réflexion collective ayant pour objet d'aboutir à une solution pour pallier à cette injustice. Merci, monsieur le rapporteur. c'est évidemment une question importante et qui qui mérite discussion la question de la déconjugalisation des prestations sociales en général est une question qui se posera et qui se pose de plus en plus souvent, il y a d'ailleurs une avancée marquée par le Sénat, l'initiative de Philippe mouiller sur la déconjugalisation de de la hache mais là il s'agit d'une demande de rapport et donc fidèle à la jurisprudence du Sénat, ce sera un avis défavorable je vous remercie.

que le plafond de ressources pris en compte pour le foyer pour le bénéfice de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant correspondent au plafond applicable ou. Couples bi-actifs cette préoccupation rejoint la question plus large des modalités de prise en compte des revenus de remplacement dans les ressources prises en compte pour le bénéfice des prestations familiales, c'est un sujet qui est évidemment important et auquel j'accorde beaucoup d'importance, mais il ne semble pas opportun de le traiter de manière isolée et surtout dans des délais aussi contraints particulier au regard de tous les chantiers qu'on a aujourd'hui apporter en matière de modernisation de notre système de de prestations sociales, je pense notamment à la question de la solidarité à la source, et je vous propose ainsi aussi de de retirer votre amendement. Merci monsieur et la comédie il est retiré de 737 est retiré le on passe aux 37 bis, une prise de parole de monsieur Iacovelli. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cette près cet article prévoit un rapport donc on connaît déjà le résultat mais je voudrais juste qu'on s'attarde un instant sur son objet. Il prévoit spécifiquement d'étudier la santé et la prévention des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. La santé, et notamment la santé mentale des enfants qui sont placés est un enjeu majeur, il est nécessaire qu'ils soient accompagnés dès leur plus jeune âge, pour assurer que chacun d'entre eux malgré leurs blessures passées puissent avoir un avenir rempli de possibilités d'opportunités de rêve, comme nous le souhaitons pour tous les enfants de France et d'ailleurs le 1er séminaire de recherche de l'eau ANPE avait lieu en mars 2021 et avait comme sujet la santé mentale des jeunes placés lors de ce dernier plusieurs chiffres ont été rappelés, chers collègues, je vous invite à aller écouter près les enfants placés, ça représente 2 % de la population de moins de 21 ans, et pourtant 25 % des sans-abri 20 pour 100 des détenus ont été confiées et ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, et je ne parle même pas de ceux qui dans des actes terroristes ont frappé notre pays et dans certaines régions, ils représentent plus de 50 % des malades d'hôpitaux de jour après une recherche réalisée par des sur des enfants placés des Bouches-du-Rhône, la prévalence des troubles anxieux et des troubles psychotiques chez ses enfants, a été multiplié par 5 pour les troubles anxieux et près de 40 pour les troubles pour les troubles psychotiques par rapport aux adolescents de la population générale c'est chiffre chers collègues doivent nous alerter le rapport proposé donc essentiel car peu d'analyse nous permettent d'avoir une image claire de la réalité des choses et c'est uniquement avec une telle vision de l'ampleur du phénomène et des besoins de ses enfants, que nous pourrons mettre en place des dispositifs ciblés certains existent déjà et ont fait déjà leurs preuves Monsieur le Ministre, je pense au programme Pégase, que nous avions étudié et souhaitions étendre par une expérimentation qui malheureusement a été déclarée irrecevable

nous sommes plusieurs à avoir déposé une proposition de loi sur la création d'une délégation aux droits de l'enfant, je pense que ça sera l'occasion de pouvoir mettre en place ces dispositifs et étudier réellement. La situation merci, cher collègue, l'amendement 100, hein, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, il s'agit à nouveau d'une suppression de d'un d'un article, bien évidemment, la question d'un bilan de santé à l'entrée des enfants dans le dispositif de protection de l'enfance et et pertinent fidèle à la jurisprudence du Sénat, ce sera un avis défavorable pour la demande de rapport, je vous remercie. J'ai dit, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le. Notamment le le sénateur Iacovelli comme vous, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, néanmoins plusieurs expérimentations sont en cours pour permettre un accompagnement beaucoup plus développé des enfants protégés, notamment sur le plan sanitaire à partir d'un bilan de santé complet des enfants dès leur prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance certaines expérimentations prenne fin mi-2023 avec un objectif de déploiement sur l'ensemble du territoire, elles feront dans ce cadre, l'objet d'une évaluation donc il me semble-t-il, permet de répondre au moins partiellement, votre votre souhait donc, comme pour les autres rapports ce sera sagesse pour le gouvernement. Merci donc je mais aux voix l'amendement 101 de la commission avec qu'un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté l'article être supprimés, nous passons à l'amendement 458 Madame Mellow. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pendant plus de 50 ans notre politique familiale a reposé sur le principe de l'universalité, cela signifie que s'adresser à tous les Français, sans distinction sociale, or ce principe d'universalité a été mise à mal, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres, cet amendement vise à réaffirmer l'universalité des allocations familiales et à favoriser la natalité Oui alors bien évidemment sur le fond, nous partageons les observations qui viennent d'être exprimées, j'ai d'ailleurs été l'auteur d'une PPL sur ce sujet qui a été votée par le Sénat, à l'évidence, la politique familiale n'est pas une politique sociale à l'évidence, je voudrais revenir sur cette modulation, mais ceux-ci posé cet amendement ne le permet pas, hein, puisque on a cherché tous les moyens de déposer un amendement, mais il serait article 40 et donc au fond ce ça revient à faire une déclaration d'intention et d'intention et et c'est la raison pour laquelle, pas du tout sur le fond, mais parce que ça n'est pas praticable, ça ne vole pas, comme on dit, ce sera un avis défavorable je vous remercie. Monsieur ministre-président mesdames et messieurs les laisser là. Madame la la sénatrice, je sais que c'est un sujet qui est souvent débattu dans cet hémicycle et mes réponses ne diffère pas et ne seront pas différente de celle de mes prédécesseurs, les allocations familiales sont déjà universel puisqu'elles sont versées à toutes les familles ayant au moins 2 enfants, la modulation des des allocations n'a pas remis en cause le principe d'universalité, je ne crois pas qu'il soit choquant que les 10 % des familles les plus aisées perçoivent des allocations d'un montant d'un montant moins élevé que les familles modestes ou moyennes. Et pour ma part, je pense que la politique familiale que nous conduisons peut à la fois avoir un objectif de natalité mais également un objectif social et c'est ce que nous portons dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 merci. Si donc je, je, mais aux voix l'amendement 458 Madame Mellow je vais le retirer

la loi de juillet 2020, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole en France et dans les outre-mer permet évidemment une amélioration des conditions de vie tout simplement des personnes concernées, avec ses 85 % du SMIC aujourd'hui, on constate que ça exclut certains certaines personnes qui devraient être concernés parce qu'ils sont, Alors, ils sont contraints de de. Il en fait il s'ils bénéficient d'une retraite à taux plein, il n'en bénéficient pas, voilà donc cette condition des assurés, percevant une retraite à taux plein, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions requises, alors il s'agit de prendre en compte cette situation pour améliorer également les personnes concernées merci. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur. Oui merci, cet amendement prévoit la remise au Parlement d'un rapport étudiant l'extension aux personnes ayant le statut de travailleur handicapé du complément différentiel de points de retraite complémentaire qui permet de porter la pension d'un exploitant agricole retraités ayant accompli l'ensemble de sa carrière en cette qualité à 85 % du SMIC, conformément à la pratique du Sénat, donc j'émets un avis défavorable à cet amendement, puisque c'est un rapport mais en même temps je me retourne vers vous, Monsieur le Ministre, pour demander au gouvernement des précisions sur les conditions d'accès à ce complément des retraités ayant bénéficié d'un départ en retraite anticipée au titre du handicap. Merci, Monsieur le le président, mesdames et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice et monsieur le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette demande de, de, de rapport parce que nous pensons qu'il n'a pas sa place dans en loi de financement de la Sécurité sociale parce qu'il s'agit d'un régime complémentaire et puis surtout, comme vous le savez, nous avons ouvert, le gouvernement a ouvert une série de concertations 3ème cycle d'ailleurs interviendra le 28 novembre prochain et donc nous renvoyons plutôt cette question à cette. Grande concertation sur les retraites, je répondrais à monsieur le rapporteur, dès que j'aurai la réponse précise sur ce à sa question. Là dessus. Merci, monsieur le Ministre, dont je mets aux voix l'amendement 427 avec 2 avis défavorable qui est pour.

Merci monsieur le président, les lois Chassaigne un et 2 ont permis la revalorisation de nombreuses pensions agricoles, ce qui est évidemment un progrès incontestable, toutefois il y a encore trop d'acteurs de la production agricole avec une pension en en dessous du minimum vieillesse de 906 euros 81 par mois, cela est vrai en particulier pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux qui ont été exclus du dispositif. Prévue par la loi Chassaigne de, c'est pourquoi il faut aller plus loin et permettra à l'ensemble des non-salariés agricoles de bénéficier d'un niveau de pension au moins égal à 85 % du SMIC, pour ce faire, nous demandons au gouvernement un rapport portant sur les conditions d'un élargissement du nombre de des bénéficiaires aux mesures de revalorisation, avec la suppression des dispositifs d'écrêtement sur les conditions d'exclusion du calcul du plafond des majorations pour enfants, ainsi que sur la prise en compte des pensions de réversion des aides familiaux et conjoints collaborateurs dans le calcul du plafond d'écrêtement, il est plus qu'urgent de garantir des conditions plus digne à l'ensemble de la profession agricole, je vous remercie. Oui, notre collègue pose un sujet intéressant et oh combien important qui la retraite agricole et des conjoints collaborateurs et aides familiaux, je pense qu'il va y avoir des discussions avec les par ce sociaux, il ne faut pas oublier cette catégorie de, de personnes bien sûr si tu demandes de rapport, donc je donnerai un avis défavorable et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter d'un certain nombre de mesures de solidarité lors des discussions sur la réforme, si elle vient un jour des retraites. Merci, monsieur le Ministre. D'étudier les conditions d'un élargissement des mesures de revalorisation, donc des pensions des agriculteurs, le gouvernement est extrêmement sensible à la situation des agriculteurs retraités notamment ceux percevant des niveaux les plus faibles de retraite les lois adoptées en juillet 2020 et décembre 2021 sous l'impulsion du président Chassaigne et à l'unanimité par les membres du Parlement ont contribué à revaloriser substantiellement la pension des retraités agricoles les plus fragiles, la pension des exploitants agricoles a été porté à 85 % du SMIC Net pour une carrière complète les cons joindre collaboratrices ont bénéficié d'une revalorisation de pension mensuelle significative au total ce sont 338600 personnes soit 30 % des retraités de droit direct du régime des exploitants agricoles, qui ont bénéficié d'au moins d'une des deux mesures de revalorisation, avec un gain moyen de 100 euros par mois, le sujet des minima de pension, fait l'objet de concertations spécifiques par le ministre du Travail actuellement avec les partenaires sociaux dont la FNSEA dont dans le cadre de la future réforme des retraites ainsi que le dédié à l'équité et la justice sociale débutera d'ailleurs la semaine du 14 novembre dans ce contexte un rapport spécifique sur les pensions agricoles ne semblent pas adaptées et donc avis défavorable du gouvernement. Avis défavorable, donc je mais aux voix l'amendement 800 pardon Monsieur Mounier. Merci monsieur le président, je profite de cet, de cet amendement pour prendre pour une prise de parole qui vous concerne, monsieur le Ministre, car j'essaie, avoir des précisions quant à l'effectivité de la revalorisation des pochoirs école otite de l'application de la loi Chassaigne dont les bénéficiaires sont également des élus locaux, notamment des maires la lettre interministérielle adresse en mars dernier aux administrations concernées, il y a Comtech la CNAV, la MSA indique clairement qu'il convient, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas jaunir compte durant leur mandat des droits en constitution à l'Ircantec pour les élus locaux, les élus locaux peuvent ainsi conserver leur mandat local et voir leurs pensions agricoles revaloriser malheureusement sur le terrain, j'ai rencontré des élus qui n'en bénéficient toujours pas, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous assurer que tous les retraités concernés, y compris des élus Véro, leur situation améliorée au plus vite.

puisqu'on a annoncé une revalorisation des retraites agricoles, or ce n'est pas le cas, ce qui a été revalorisé c'est le plancher mais le seuil minimum retraités de l'agriculture ne doit pas percevoir moins de 85 % du SMIC, or il y en a, bien souvent, qui avait des situations vraiment difficiles qui ont cumulé emplois et puis ben quand on on solde toutes les retraites s'ils arrivent à 85 % du SMIC on remonte pas leurs retraites agricoles, donc il y en a beaucoup qui sont arrivés en disant mais on comprend pas, on nous avait annoncé que notre retraite agricole allait augmenter, or ce n'est pas le cas, donc il y a déjà une ambiguïté sur la présentation il y a beaucoup de frustration dans les territoires, il faut non seulement faire de la pédagogie, mais en plus considérer que c'est pas parce qu'on est un agriculteur qu'on doit avoir quatre pourquoi 85 C'est ça, salaire minimum garanti, donc voilà, il faut vraiment revoir dans la pendant la réforme des retraites, la situation des retraités de l'agriculture de leur conjoint, et puis aussi des commerçants, des artisans, évidemment ils ne sont pas les seuls, mais là il y a une vraiment une incompréhension sur ce qui s'est passé le jour même. Merci, monsieur le Ministre. Oui, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, pour répondre à Madame la sénatrice, hein, je l'ai dit, c'est une, c'est une question sensible à laquelle on sera particulièrement vigilant dans les concertations qui qui s'ouvre, l'objet de mon propos était plutôt de montrer les faits justement des précédentes mesures pour répondre au rapporteur mouillé, vous dire que cette mesure a bien été inscrite dans la loi, notamment dans la loi, pouvoir d'achat de de cet été, donc les, les, les élus sont bien inclus maintenant dans ces mesures et que, à l'article 44, terre de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, vous avez une extension de la mesure aux élus des chambres agricoles,

Merci monsieur le ministre. Faut donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement 800 avec 2 avis défavorables, donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par indique cinquante-six le scrutin est ouvert.

résultat du scrutin pour cet amendement 801 Votants 329 329 pour 92 contre 237 le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à l'amendement 100 de monsieur le rapporteur. donc mes chers collègues, du fait du vieillissement démographique à l'oeuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail et ce chaque année dans ce contexte particulier, la France est appelé à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite, les partenaires sociaux sont aujourd'hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives, en ce qui concerne la place des seniors dans notre société à l'heure où l'allongement de la durée des carrières à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse face à l'urgence de la situation, cet amendement institut une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de traites, réunissant des représentants des partenaires sociaux de l'état des associations familiales, des retraités, ainsi que des personnalités qualifiées, peut être du monde agricole et l'achat et la charge cette commission de proposer des mesures, à savoir mesures favorisant le maintien des seniors dans l'emploi mesures garantissant la prise en compte de la pénibilité au travail du handicap des carrières longues dans la définition des conditions d'ouverture et de calcul des droits à pension et d'accès aux minima de pension ainsi que pour l'aménagement du temps de travail, des mesures harmonisant les règles d'attribution des pensions de réversion une majoration des pensions pour enfants entre les régimes obligatoires de base des mesures tendant ta tête à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et permettant de ramener la branche vieillesse à l'équilibre d'ici 10 ans ces préconisations ferait alors l'objet d'un projet de loi ou de dispositions spécifiques du Plfss pour 2000 vingt-quatre et serait débattu par le Parlement dans le cas où la convention n'aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétrique serait appliqué à compter du 1er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter ainsi aux générations futures d'autres devoir travailler au-delà de 65 ans, ces mesures seraient le maintien de l'âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans, ce n'est pas inscrit dans la loi actuellement l'accélération de la mise en oeuvre de la réforme Touraine de 2014 qui porte, je rappelle la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 73, nous proposons la génération 1967 pour ouvrir cette pardon progressif de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération là aussi 1000 et la convergence des régimes spéciaux vers paramètres avant 2033 selon des quand le des conditions et un calendrier, a fixé par décret en Conseil d'État. Mais c'est le président, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le le rapporteur. Alors, vous faites preuve d'une très grande cohérence d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale à l'autre en portant en portant un amendement sur le recul de l'âge de départ à la retraite, la discussion de cet amendement intervient cette année dans un contexte que nous avons déjà évoqué, qui est très particulier, puisque mon collègue Olivier Dussopt est en pleine concertation actuellement sur les différents sujets que vous mentionnez dans votre amendement, nous nous rejoignons sur les objectifs et sur les thèmes qui figurent dans votre proposition, travailler plus longtemps pour assurer l'équilibre, notre système de retraite agir en faveur de l'emploi des seniors et de la justice sociale, mieux prendre en compte les carrières longues et difficiles, mais nous avons fait le choix de la concertation et d'un projet de loi en janvier, pas d'une mesure dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale, nous ne pouvons préempter les décisions sans avoir conduit ces discussions, nous voulons respecter l'engagement que nous avons pris avec les partenaires sociaux pour conduire les trois cycles de discussions sur l'emploi des seniors il usure professionnelle sur l'équité et la justice sociale, mais également sur l'équilibre du système de retraite cycle qui s'ouvrira comme je l'ai dit tout à l'heure, le 28 novembre prochain la première ministre a également invité l'ensemble des groupes parlementaires à faire part de leurs propositions, en les invitant à un dialogue préalable aux dépens au dépôt d'un projet de loi elle réuni avec Olivier Dussopt, tous les présidents de groupe en ce sens, Olivier Dussopt a poursuivi d'ailleurs cette semaine l'ensemble de ces échanges, alors, n'anticipons pas les débats que nous aurons prochainement, laissons la place aux concertations préalables sans cranté des dispositions dans la loi, pour cette raison, le gouvernement demande le retrait de cet amendement. Merci monsieur le ministre, monsieur Iacovelli. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, encore une fois, je pense que nous nous sommes tous favorables sur les bancs de de cette assemblée à une réforme des retraites. On n'a pas toutes tous les mêmes solutions en l'occurrence, on a entendu lors des concertations

ont lieu en 3 Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé les partenaires sociaux sont tous présents, même la CGT revient à la table des discussions pour vous dire que les choses avancent, d'ailleurs, nous avons tous été en tous les groupes ont été représentés cette semaine pour les discussions lors du cycle, les comptes rendus du cycle numéro un tous les groupes sauf chers collègues Les LR les républicains, vous avez refusé de participer à ces consultations et à ces discussions pour pouvoir avancer sur un projet, un projet de loi donc vous oui mais ça fait six ans vous faites un marronnier avec un amendement, je pense que toutes les oppositions était favorable à un vrai texte de loi sur la réforme des retraites et ne pas passer par un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale, donc vous comprendrez bien que même si nous sommes favorables à une réforme des retraites, nous ne pouvons pas être favorable à passer à un passage par amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale et c'est pour ça que le groupe RDPI, votera contre cet amendement.

René-Paul Savary montre la constance de la majorité sénatoriale et montre aussi son opiniâtreté pour défendre un projet qui est cohérent avec la trajectoire qui nous est aujourd'hui montré sur la branche vieillesse, le déficit est tellement important et de tellement de plus en plus important qu'il faudra bien prendre des mesures, sinon si nous les prenons pas c'est les générations d'après qui seront obligés de prendre leur retraite beaucoup plus tard, bien sûr vous avez entamé des des travaux, mais n'oublions pas qu'il a eu aussi 3 ans de travaux auparavant il faut il faut s'en inspirer, que nous avons des éléments en tout cas moi je voulais insister sur un premier principe, c'est d'abord donner vraiment sa chance à la négociation entre toutes les parties prenantes, parce que ce que propose René-Paul Savary, c'est évidemment une plus qu'une conférence est désormais une convention nationale qui pourrait prendre le temps puisqu'il donne un an aux partenaires sociaux à se décider sur l'emploi des seniors sur un certain nombre de sujets comme les retraites de réversion sur les les difficultés des emplois qui sont, qui sont, comment un un peu difficile et qui finalement font que les personnes sont plus tôt à la retraite en difficulté donc il y a un certain nombre de sujets et et qu'il faut absolument débattre le second principe cette définir nous-mêmes les paramètres qui nous semblent les plus pertinents pour atteindre cet équilibre parce que ces paramètres sont forcément financier car nous débattons d'un PLFSS ils sont à la fois une feuille de route pour les partenaires sociaux qui donnent l'ampleur des mesures d'équilibre qu'il convient de négocier et un cadre surtout normatif ayant vocation à s'appliquer à compter de 2024 en cas d'échec après 4 ans de rejet de ses propositions et alors que vos projections du chef font craindre de lourds déficits, il est temps d'agir. Merci, cher collègue Monsieur Wagner Arenberg. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je le rapporteur, je suis d'accord avec René-Paul il le c'est sur le fond, parce qu'il faut une réforme je crois que ce qui le ni ni aussi la réalité qui est dans tous les rapports évidemment et notamment celui du corps qu'il faut réduire les inégalités, aussi il faut réduire je dirai les déficits, il y a 12 milliards de prévus en 2000 26 2027 180 milliards en 2035 si on les cumule donc il faut agir, je ne reviens pas sur la réduction des inégalités, tout a été dit j'insisterai simplement sur le un point sur la, le maintien des seniors en activité, qu'on soit 56 en moyenne actuellement entre les 55 64 ans, très très inférieur à la moyenne de l'OCDE, qui est de 66 ans, il y a donc un progrès nécessaires à opérer pour travailler un peu plus longtemps, donc il faut aussi que cette réforme soit acceptée socialement et politiquement. C'est ça le point essentiel, parce que sinon effectivement, on sera à la merci, effectivement, de revenir à la faveur d'une autre majorité, ce que je ne souhaite pas, mais sur cette réforme, j'ai participé, je regrette que certains n'y soit pas à à la conférence, enfin disons au bilan d'étape que nous a donnée monsieur Dussopt, c'était très intéressant, on voit qu'il y a des convergences pour réduire ces inégalités restent effectivement les mesures techniques, je dirais à prendre, il y a des solutions acceptables, je crois que aujourd'hui on part à la retraite environ à 62 ans et demi, pourquoi ne pas atteindre plus facilement et plus rapidement sans aller jusqu'à 64 ans, les 63 ans, et puis pourquoi ne pas accélérer aussi la réforme Touraine voilà, moi je pense que il faut maintenir quelque chose d'acceptable, parce que je crois beaucoup, il fera l'acceptation et au paritarisme et donc pour toutes ces raisons, parce que je crois qu'on on va un peu loin

Il y a beaucoup de raisons pour s'opposer à cet amendement mais je prendre un seul point en France. En moyenne, il s'écoule 2 ans entre la cessation d'activité, la retraite et les ouvriers, les employés ont un écart bien supérieur à 61 ans, ils ne sont plus que 28 % d'emplois, une partie des autres sont au chômage, mais ils seront moins nombreux et moins longtemps le gouvernement. Et la droite, ils ont veillé, d'autres sont en avait mais aucun progrès n'a, n'est à tu n'es attendre car le patronat ne veut pas entendre parler de pénibilité physique ni d'usure psychique et la France reste le mauvais élève en sinistralité, d'autres enfin sont restés au RSA mais la prochaine veut réforme va s'en occuper, une personne sur 3 dans cette situation, ni en emploi ni en retraite est en dessous du seuil de pauvreté, et ils y resteront, grâce à vous, de plus l'espérance de vie des hommes ouvriers étant inférieur à 6 ans à celle des cadres et de bien plus quant à leur espérance de vie en bonne santé, si le Sénat adopte cet amendement il participera écrire une des pages les plus inégalitaires sur le plan social, rien ne justifie l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite et notamment tant que n'est pas réduit massivement l'écart entre l'âge de l'exclusion de l'emploi et l'âge légal de départ et d'autant que la durée du temps de vie à la retraite diminue déjà que les gains d'espérance de vie ont été versés au travail par les réformes précédentes et qu'une grande partie des Français modestes n'arrive plus à la retraite en bonne santé, car si pour 25 % des 10 % les plus pauvres, ceux-là reste la retraite des morts pour beaucoup, c'est encore la retraite avec incapacité nous nous opposons donc à cet amendement. Merci, cher collègue Madame Lubin. Merci monsieur le président, nous reconnaissons effectivement la constance de notre collègue René-Paul Savary, qui propose chaque année, cet amendement et cette année il a assorti donc d'une d'une demande de de de concertation élargie au travers d'une d'une convention, je pense, de manière à ce que ça soit un peu moins abrupt que d'habitude, compte tenu du fait qu'il est quand même un grand défenseur du paritarisme, tout comme nous, et que donc adopter une un tel amendement comme ça à la va-vite un PLFSS pouvait paraître quand même un, un petit peu curieux, bon, nous nous sommes opposés sur le fond, vous le savez, ça ne surprendra personne, nous espérons qu'il y aura un débat puisque de toute façon, il faut bien se rendre à l'évidence, le gouvernement a l'intention de reculer l'âge de départ à la retraite, il y aura donc un débat, nous l'espérons et nous développerons nos arguments en cours de débats mais rapidement, nous y sommes opposés, déjà parce que c'est une retraite qui sera d'une injustice incroyable, l'objectif sera de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, enfin dans les caisses de retraite pardon immédiatement, et donc il faudra clairement empêché de partir ceux qui sont près de l'âge de la retraite de, de, de, de les empêcher de valider leurs droits à la retraite et ça touchera des gens qui travaillent depuis longtemps, qui ont les métiers les plus difficiles, enfin vous connaissez vous le savez, tout ça aussi bien que moi, ensuite je ne vraiment je ne peux pas, je ne peux pas laisser dire laisser faire ses discours alarmiste, le corps effectivement fait état de déficit sur les 5 ou 6 ans qui viennent, qui sont loin d'ailleurs, il faut lire le rapport du COR élire les conclusions qui sont loin d'être aussi alarmistes que ce que l'on peut entendre et faire croire aux Français que si on ne fait pas de réforme dans les mois qui viennent, mais paraît en péril notre système de retraite, c'est leur raconter des histoires, la suite au prochain numéro. Merci, cher collègue Monsieur lévrier. Merci monsieur le président, de choses sur la forme, d'abord je je je loue la constance mais parfois à géométrie variable de notre rapporteur, René-Paul Savary parce qu'effectivement, tous les ans depuis 5 ans, il revient par un amendement sur le système de retraites en revanche et ça rejoint le fond maintenant sur la façon de faire, là, il demande une négociation négociation que ne suivent pas l'air d'un côté, négociations qui est déjà engagé, pourquoi demander quelque chose qui existe déjà, puisque c'est en cours, c'est mon 1er point et le 2ème point qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que le PLFSS traite des paramètres d'équilibres financiers. Notre système de retraite n'est pas que ça, notre système de retraite sa vraie valeur, c'est son c'est sa logique intergénérationnel, c'est ça, c'est sa solidarité, c'est le fait que les actifs financent la retraite des personnes en retraite et là on en parle pas, à travers un PLFSS on ne peut pas en parler et on a bien vu depuis ces 5 ans où il y a une une approche tout à fait différente qui a voulu être fait et qui, qui n'a pas pu se faire à cause de la Covid, je vous le rappelle, de toutes les inéquités qui existe dans le système de retraite 40 de caisse de retraite des inédite qui était incroyable sur un nombre de points incroyable, et quand on parle de financement, certes, le coeur n'est pas aussi alarmistes que certains veulent le dire, mais il le devient si on veut réduire ses inéquité si on veut parler des réversion qui ne sont pas comme il faut, si on veut parler des de l'égalité femmes-hommes à travers la retraite et ainsi de suite, je pourrais prendre un certain nombre d'exemples, donc oui il faut une réforme, oui il faut de la concertation, mais certainement pas à travers un PLFSS

Merci monsieur le président, dans un 1er temps, le président de la République avait annoncé l'allongement de la du départ à la retraite par voie d'amendement dans le PLFSS 2023 face à l'opposition unanime des organisations syndicales et de certaines organisations d'ailleurs patronale, le gouvernement a reculé entamé une série de concertations ayant pour objectif de présenter un projet de loi spécifique à la rentrée 2023 c'est dans ce contexte, pour la 4ème année consécutive que notre collègue René-Paul Savary propose cet amendement pour réformer le système des retraites oui on peut le dire, il est constant, la version 2022 prévoit de mettre en place dans un 1er temps une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites qui doit établir des propositions pour garantir l'équilibre du système de retraite dans ça se comptant l'amendement prévoit qu'en cas de désaccord des mesures paramétrique seraient mises en place, il s'agit d'un cocktail explosif de 4 mesures régressives premièrement le report progressif de l'âge de départ à la retraite à 64 ans pour la génération 67, deuxièmement, la suppression de la décote à 67 ans, troisièmement l'accélération du calendrier de la loi Touraine à 43 annuités pour la génération 67 au lieu de 73, quatrièmement, la suppression des régimes spéciaux Les LR n'était pas là à la table de monsieur Dussopt pour discuter du projet de réforme des retraites, car finalement vous partagez la même philosophie, je répondrai ple ment sur l'argument de la sauvegarde du système de retraite, le dernier rapport du conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit temporaire entre 22 entre 2022 à 2032 du régime de retraite ayant de retrouver l'équilibre, il n'y a donc pas de danger sur l'avenir du système, d'autre part, les salariés et les retraités ne sont pas responsables de ses déficits, mais des politiques successives qui ont entraîné des mesures d'économies sur la masse salariale. Je vous remercie, Merci la promotion de notre collègue Savary au nom de l'équilibre du régime des retraites, ce n'est pas une première, ça a été dit, c'est une constante, mais c'est aussi un recul social considérable pour l'ensemble des salariés, comme l'a rappelé ma collègue Katia pour se polie mais en particulier, moi je vais me concentrer sur les femmes, vous le savez, actuellement, les femmes sont pénalisés dans leur carrière est à la retraite par des pensions inférieures aux hommes pour des carrières équivalente pour les femmes, l'allongement de la durée de cotisation, le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est la double peine, elle qui touche en moyenne 25 % de salaire en moins que leurs collègues masculins à poste égal, et qui ont des carrières courtes ou haché doivent déjà partir en retraite plus tard d'un an en moyenne que les hommes et leurs tensions sont elles aussi en moyenne plus faibles de 42 cet amendement va aggraver cette situation, renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes, si l'objectif est véritablement de réduire les déficits, il y a une solution très simple qu'on vous propose à chaque fois que que vous refusez, augmenter les recettes, plutôt que de réduire les dépenses, relancer l'emploi public, y compris des seniors réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et, enfin, augmenter les cotisations pour résoudre le déficit qui est prévu par le corps en 2027, il suffirait d'augmenter de 4 euros 50 le salaire mensuel à partir de 2023 et même en envisageant de ne pas accabler les : les patrons de couper la poire en 2, et de l'augmenter de 2 euros 50 en plus pour les cotisations employeurs et 2 euros pour les cotisations salariés vous avez résolu le problème du déficit du système de retraite donc mes chers collègues, et Monsieur le Ministre, plutôt que d'aggraver les inégalités dans notre pays et de faire travailler les les salariés toujours plus longtemps, commencer par utiliser le levier efficace économiquement et socialement.

vous parliez de telle heure de méthode et de participation aux différentes réunions, au groupe de travail ben notre méthode, vous l'avez vous l'avez par cet amendement, vous connaissez notre position aujourd'hui à partir de notre position, nous sommes prêts à discuter, mais nous avions besoin de se mais ce message politique pour dire clairement où nous voulons aller et pourquoi nous voulons le faire et cet amendement est un point essentiel : nous faisons pas d'illusions, le 3 aura forcément une intervention et donc sur cet amendement, mais au moins nous avons le mérite ici au Sénat d'être cohérents dans notre démarche d'avoir des solutions à apporter, qu'elle plaise ou qu'elle déplaise mais en tous les cas, d'avoir une vraie responsabilité sur cet enjeu fondamental pour maintenir à la fois notre système de retraite, les niveaux de pension et surtout corriger des inégalités et en matière d'égalité, je voudrais revenir sur une proposition du groupe LR qui n'a pu être rédigé, étant donné la la l'article, mais qui concernent notamment les parents qui ont des enfants handicapés, pour lequel nous souhaitons réellement faire évoluer les choses pour que les pensions de réversion du dernier survivant puis serait reversée aux enfants handicapés à l'issue notamment malheureusement au moment du décès du parent, c'est pour nous un élément, un exemple de justice sociale, sur lequel nous souhaitons clairement intervenir et Monsieur, c'était un message de par vos fonctions, nous étions à porter et puis pour terminer en matière de méthode, je voudrais simplement dire que nous appuyons sur des outils existants, la réforme Touraine je veux, j'ai repris les arguments à l'époque de la réforme Touraine qui était un une évolution sur lesquels nous nous appuyons pour apporter aujourd'hui des éléments importants, et donc je me souviens des interventions du groupe socialiste à l'époque et je voudrais surtout dire hein messieurs lévriers a communique en matière de méthode lorsqu'on voit la méthode ne donne sera mis Delevoye je pense qu'à partir de là, vous pouvez avoir un peu plus d'humidité sur la façon de faire. Merci, cher collègue Monsieur Milon. merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, en en vous écoutant, je me suis peu interrogé sur certaines choses, vous avez dit qu'il fallait faire une concertation et dans le cas du 1er mandat du président de la République, hein Monsieur Monsieur Delevoye avait été nommé commissaire du gouvernement, et il nous a dit on a auditionné X fois avec René-Paul Savary, qu'il l'avait fait des négociations et qu'il avait apporté un rapport au président de la République est-ce que finalement ce monsieur, commissaire du gouvernement, donc recevoir un salaire au moins égal à celui d'un ministre a été payé pour rien, deuxièmement, je voudrais revenir sur les les négociations à ce que avec Monsieur Savary dans le cas des commissions d'affaires sociales nous avons nous aussi auditionné les syndicats nous avons auditionné le patronat sous là ou pas, sous le haut patronage de Gérard Larché, nous avons organisé de conférence nationale présidée par le 1er ministre Édouard Philippe qui, à chaque fois, a confirmé la nécessité de réformer les retraites, a confirmé la nomination de Monsieur Delevoye et a confirmé le rapport de monsieur Delevoye, donc nous sommes dans dans ce cas-là. Normalement on bien en droit de pouvoir faire des propositions après négociations un accord du 1er ministre et après une négociation et concertation avec le commissaire du gouvernement chargé des retraites, certains reprochent ou constate sous forme de reproches, la constance de Monsieur Savary c'est une constance, ça n'est pas un entêtement c'est une constance, il a même amélioré ses propositions, elles sortent des négociations que nous avons eu avec les syndicats avec le patronat avec le 1er ministre et avec le commissaire au gouvernement. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que le le groupe les indépendants a toujours été favorable à une réforme des retraites, ceci étant dit, je voudrais aussi vous vous faut rassurer sur le fait que nous sommes favorables à cet amendement sur le fond, mais cette année, la situation est complètement différente de celle que nous avons vécu l'année dernière, la réforme est en cours, les prémices de la réforme sont en cours, j'ai assisté la semaine dernière au nom du groupe à la réunion au ministère du Travail, le bilan qui a été dressé était très voilà très très à ce ce qui peut être souhaitable et la concertation des partenaires sociaux, a commencé, enfin les les choses vont dans le sens souhaité, donc nous devons semble-t-il attendre que l'examen du projet de loi nous arrive et il n'est pas raisonnable de de voter, nous semble-t-il favorablement cet amendement, c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous y opposer, nous nous abstiendrons à la quasi-unanimité. Merci Monsieur Viénot. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est Michel Rocard qui disait que la réforme des retraites je crois ferait tomber plus d'un gouvernement, alors je ne sais pas si c'est vrai tomber mais j'aimerais en tout état de cause, hein, il y a eu la réforme Balladur de 93, les 40 ans de cotisations en 2003 le recul d'âge de la retraite à 62 ans en 2010 et la réforme tourisme Touraine en 2013, qui n'est pas la moindre des. Des réformes, je pense que le pays il y a une forme de de nostalgie par rapport à la retraite à 60 ans, pas faut pas cacher cette réalité, mais la nostalgie, ça ne fait pas bonne politique il y a une évidence, c'est qu'il y a besoin dans ce pays d'une réforme des retraites, et moi je ne partage pas ce que vous avez dit monsieur Martin lévrier la réforme des retraites, la dernière fois, elle a échoué, mais pas seulement à cause du Covid elle a échoué parce que à la fin on savait plus si elle était systémique si elle était paramétré qui est parce que il y avait un désaccord sur le fond au plus haut lieu disons les choses telles qu'elles sont : le Covid a eu bon dos sur cette question, mais la réforme des retraites, c'est simple, c'est toujours trop tôt, c'est toujours trop tard, problème de forme, et bref il faut jamais l'affaire, or je pense que c'est un question une question centrale pour notre pays, j'ai été sensible autrefois une argumentation de notre collègue Jomier en constatant que les prélèvements obligatoires étaient très élevés dans notre pays mais que, au fond, ces prélèvements obligatoires, il était très élevé, mais qu'on se consacrer assez peu de moyens à l'investissement et au fonctionnement des services publics, hé bien c'est juste et pourquoi, parce qu'on redistribue beaucoup vu redistribue énormément, et donc la question c'est : c'est d'avoir des réformes qui fasse que on maîtrise la redistribution qu'on arrête d'ailleurs l'échec de ceux-ci, l'échec de ceux-là, même s'il y a toujours des bonnes raisons de le faire et qu'on soit en capacité par rapport au à l'argent qu'on prélève, je ne crois pas qu'on peut augmenter les recettes et bien d'avoir une politique cohérente et d'avoir une capacité d'investissement pour l'avenir des services publics et de faire fonctionner ses services publics correctement, je pense que c'est ça l'avenir de notre pays, je vous remercie. Merci, cher collègue, le Sofia l'air. Merci monsieur le Président, on savait que cette question serait sensible, c'est vrai que toutes ces années, on n'a pas voté le l'amendement, le groupe RDSE, l'amendement ça varie parce qu'on pense que ces réformes de retraites doivent pas passer par un amendement en PLFSS en revanche, cette année, les choses étaient un peu différentes puisque on a eu quand même une campagne présidentielle avec un président qui a mis ouvertement sur le le chantier cette réforme de la retraite et d'allongement des cotisations alors moi je vais même plus loin : moi, je suis même pour la retraite par points, mais bon, il faut laisser les les partenaires sociaux se mettent d'accord, la seule particularité, aujourd'hui, c'est qu'enfin les partenaires sociaux se sont remis autour de de la table pour pouvoir renégocier et autant arriver à une réforme qui soit consensuelle partagée et responsable, je crois qu'il est responsable, plusieurs façons de voir les choses, travailler plus longtemps, c'est pas simplement cotiser plus longtemps pour les retraites s'est cotisé aussi pour le reste des branches de la Sécurité sociale et on sait bien que dans les années qui vont venir avec le vieillissement de la population, on aura besoin de recettes supplémentaires faut faut pas non plus mentir à aux générations qui viennent, on va voir des dépenses supplémentaires, la 2ème chose c'est que si vraiment ça provoquait des excédents importants, moi ça me dérange pas qu'on relève le montant des retraites, que je sache on nous retraités sont pas des nantis et on peut augmenter ses ses cotisations, alors nous ne voterons pas cet amendement soit compte soit en nous abstenant pour le le groupe mais en revanche on a bien entendu le message et l'année prochaine, si les choses ne sont pas réglés, je peux vous assurer qu'il en sera autrement. Oui, merci Monsieur le le président, bon moi je vais voter, bien sûr, cette avant cet amendement mais j'ai quand même une question est-ce que reculer l'âge de la retraite va suffire si on ne fait pas une vraie réforme de la famille puisque aujourd'hui il y a pas assez d'actifs, donc je pense qu'il va falloir aussi pensé à faire une vraie réforme de de la famille, voilà je vous remercie. Tout le monde est attaché au système par répartition, il ne veut pas le remettre en cause. Oui. Or si on finance notre système de répartition par la dette, on le remet en cause, donc il ne faut pas le financer par la tête, et effectivement il faut trouver des recettes. Nous savons que nous avons un système compliqué et je pense que maintenant tout le monde s'accorde à dire que, compte tenu de sa complexité, faire une réforme systémique, c'est dans notre pays impossible bouger tous ces paramètres, tous ces régimes, c'est particulièrement compliqué, donc vaut mieux se rabattre, me semble-t-il, sur une réforme paramétrique, à condition de la rendre acceptable la réalité, je crois que tout le monde la partage un an un taux de d'emploi des seniors, qui est le plus bas parmi les pays européens, on a un âge de départ à la retraite le plus bas parmi tous nos voisins tous nos voisins européens, ne l'oublions pas, on a une démographie ou le nombre de cotisants augmente mais le nombre de retraités augmente beaucoup plus vite, on a également une espérance de vie qui a augmenté en plus ou moins bonne santé, certes, mais qui a augmenté, donc il faut rééquilibrer le temps de travail et le temps de retraite c'est particulièrement nécessaire et nous avons nous émis un certain nombre de principes mais que je suis sûr beaucoup faire confiance aux partenaires sociaux, qui ne partage pas ce principe ne pas faire de retraités pauvres et le système actuel, les rapports du COR, quel que soit ce que l'on peut en penser, montre bien que on n'arrive pas à l'équilibre et en ayant un niveau moyen de vie des retraités qui sera plus bas que celui qui existe aujourd'hui et notre volonté, également, et là il y a quelques divergences, c'est de ne pas tarder à prendre des réformes et ce qui conduirait à ce que l'on travaille au-delà de 65 ans, comme ça se fait dans dans de nombreux pays européens où les gens à soixante-dix ans reprennent des petits travail pour pouvoir vivre, exemple, la Suède, nous ne souhaitons pas d'un travail au-delà de 65 ans, c'est pour ça qu'on fait un certain nombre de propositions Effectivement, Jean Marie venant d'Arenberg dit je ne souhaite pas le décalage là naturellement, naturellement, de par les réformes Touraine qui ont été prises. Naturellement, l'âge de départ augmente et va jusque 63 voire 64 ans, et la mesure en prenant à un âge qui suit justement cette tendance pour le taux plein permet véritablement d'être incitatif sur l'emploi, ce que l'on souhaite et puis également l'intérêt de pouvoir équilibrer le système tel que nous le vous, nous vous le proposons cet intérêt c'est de faire en sorte de générer quand même des recettes supplémentaires qui permettent de prendre en compte toutes les difficultés, les inégalités, toutes les mesures sociales qui doivent s'adapter au maintien des emplois dans le senior, sinon nous n'aurons pas la possibilité de prendre en compte le handicap, la maladie et un certain nombre de paramètres qui sont effectivement pénibilité et d'autres qui sont effectivement tout à fait important si on maintient les seniors en emploi, donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que notre réforme permet de répondre à toutes ces attentes légitimes que vous avez soulevés je répondrai également à à quelques intervenants, qu'il y a une différence effectivement par rapport à ce que nous pensons que le gouvernement propose puisque jusqu'à présent, c'est encore en débat, nous pensons que cette proposition fait que elle est moins brutal, un an de discussions encore avec les partenaires sociaux pour s'entendre sur un certain nombre de dispositions, donc pas d'étatisation du système telle qu'il était proposé par la réforme Delvoye, ne l'oublions pas, et puis également, nous ne souhaitons pas que l'on travaille au-delà de 65 ans, et nous ne proposons pas, je vous le rappelle, la suppression des régimes sociaux, pourquoi, parce que nous pensons.

que ce sera particulièrement difficile, il n'acceptez, c'est pas la peine, vaut mieux progressivement comme ça déjà été fait par le passé les aligner sur un régime général, ça nous paraît là aussi un moyen de faire comprendre que l'ensemble de ces paramètres peuvent être discutés de façon à arriver à faire en sorte que les générations futures reprennent confiance pour leur retraite. Si monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Monsieur le le président, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le le rapporteur Savary, vous l'avez compris je crois que le gouvernement partagent de nombreux constats avec la majorité sénatoriale, et notamment la nécessité de réformer rapidement notre régime de retraite à la fois pour en assurer l'équilibre et je sais que nous ne partageons pas manifestement la même lecture du rapport du COR, mais pourtant, elle est extrêmement elle extrêmement clair, mais également pour créer de nouveaux droits est notamment visé à ce que notre système, il soit plus égalitaire qui prenne mieux en considération la réalité des des carrières des professionnels et puis qui l'accompagne aussi la réalité, celle du vieillissement de la population. Et vous savez qu'à côté de cette réforme des retraites, je conduis avec avec nos concitoyens une concertation autour de la question du bien vieillir dans laquelle la question de l'emploi des seniors va tenir une place extrêmement importante, on partage avec vous cette nécessité, néanmoins on vous souhaiteraient aller comme vous le savez, relativement vite, puisque le président de la République a notamment annoncé qu'il souhaitait que cette réforme puisse prendre corps avant la mi-2023, tant la nécessité de de réformer est extrêmement importante et que, dans cette et qu'on essaye de concilier avec notre méthodologie la nécessité d'aller vite et en même temps, d'assurer une acceptabilité sociale et politique de cette réforme dans une concertation large donc pour laisser et être on va dire sincères dans cette concertation, on préfère ne pas cadrer en avance les termes du débat ni imaginé ou renvoyer à un atterrissage cadré de cette réforme, ce que vous proposez, dans le cadre de la concertation que vous, vous vous proposez donc c'est là la différence majeure qu'il y a entre nous deux propositions et fort quand même de ces éléments de convergence qui me semble plus important que les éléments de, de, de divergences je repropose de retirer sa peine cet amendement et de faire confiance à la concertation qui qui s'ouvre avec le gouvernement. Merci, monsieur le Ministre, j'imagine que l'amendement est maintenu. Monsieur le rapporteur. Donc j'ai été saisi oui, madame la présidente. Oui, très vite, pourquoi on a mis des mesures aussi c'est parce qu'on est un PLFSS hein, donc si on avait fait simplement un amendement de pour une convention mais ce que je voulais dire et et je réponds à ceux qui qui soutenait la précédente réforme, moi je suis un peu toujours surprise de cette histoire parce que on nous l'a présenté pendant 2 ans et demi et je me souviens de débats ici à la mi-longs là dit avec avec Jean Paul Delevoye, avec le Premier ministre, Édouard Philippe, c'était la réforme du siècle, juste, formidable qui allait tout résoudre je ne comprends pas pourquoi tout simplement, elle est toujours au Sénat, elle a été votée au 49 3 en mars 2020, pourquoi ça n'est pas celle-ci, que vous avez ressorti donc voilà c'était simplement une observation. Merci ma ma présidente, donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes républicains et CRCE sur l'amendement 102 je vous rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par article 56 de règlement, le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin sur l'amendement 100 de de la commission votants 344 exprimés 325 pour 195 contre 130 Le Sénat a adopté. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 45 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est pardon, madame la présidente. Plus d'une annonce pour les commissaires des Affaires sociales, je vous propose de vous retrouver à 14 heures 30 en salle des commissions qu'elle nous avons un amendement du gouvernement examiner. Merci madame la présidente, la séance est suspendue.